Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui les crédits de la mission « Action extérieure de l'État », qui porte la majorité des moyens du ministère des affaires étrangères, avec la mission « Aide publique au développement Le projet de loi de finances pour 2023 prévoit l'ouverture de 3,2 milliards d'euros de crédits en autorisations d'engagement comme en crédits de paiement. Ainsi, les crédits augmenteraient de 5,2 % en valeur et de 0,9 %, une fois corrigés de l'inflation. L'essentiel de la hausse des crédits s'explique par les évolutions de trois grands postes de dépense. Le premier concerne les dépenses de personnel, qui augmenteront de 64 millions d'euros cette année. évolution témoigne d'un véritable relâchement des efforts qui avaient été entrepris par le ministère ; je dirais même d'une forme de reniement au détriment de nos finances publiques. Depuis l'année dernière, le ministère s'est engagé dans une réforme des rémunérations qui se traduit par une augmentation de 30 millions d'euros, en cumulé, des mesures catégorielles. En parallèle, rien n'a véritablement été fait pour maîtriser et réformer les indemnités de résidence à l'étranger,

D'autre part, ces indemnités continuent d'être défiscalisées, ce qui n'est pas acceptable. L'État paie deux fois, en versant l'indemnité et en se privant de l'imposition sur le revenu. Enfin, le budget prévoit la création d'environ 100 équivalents temps plein, ce qui efface ainsi un tiers des efforts réalisés dans le cadre d'Action publique 2022. J'avais déjà eu l'occasion de regretter que le ministère des affaires étrangères n'aille pas au bout de la réforme Action publique 2022 et ne réalise pas l'ensemble des efforts qui lui étaient demandés. J'observe donc que, outre le fait de ne pas avoir atteint ses objectifs, le ministère les efface pour un tiers dès cette année. Cela ne contribue pas à donner crédit à la parole de l'État et du Gouvernement dans son engagement d'assainir nos finances publiques. Le deuxième poste d'évolution des dépenses concerne les contributions internationales versées par la France. Rémi Féraud et moi-même avons réalisé cette année un contrôle sur les contributions internationales versées par notre pays. Nous avons noté que la France devait prendre conscience de la perte d'influence qu'elle avait subie au cours des dernières années, faute d'investir suffisamment. En 2023, les contributions internationales augmenteront de 55 millions d'euros. J'aimerais dire que ces crédits traduisent une montée en puissance de notre participation à certaines organisations, mais la réalité est qu'il s'agit surtout de maintenir les crédits à niveau constant, compte tenu de la dépréciation de l'euro face au dollar. Nous observons en effet que la dépréciation de l'euro entraîne une augmentation de 52 millions d'euros sur les contributions versées en dollars ou en francs suisses. Cependant, nous voudrions décerner un satisfecit au ministère de l'Europe et des affaires étrangères (MEAE), qui a enclenché le mécanisme de couverture de change très tôt, permettant ainsi d'éviter d'importantes pertes de change. Celles-ci pourraient s'élever à environ 20 millions d'euros si les paiements avaient lieu dans trois mois. Enfin, les dépenses immobilières augmentent de plus de 20 millions d'euros, ce qui s'explique par les effets de l'inflation et une programmation dynamique. Il s'agit d'abord de dépenses courantes d'entretien, qui augmentent sous l'effet de la hausse des prix de l'énergie. Les dépenses d'investissement à l'étranger augmentent pour mettre en oeuvre le schéma directeur. Avec Rémi Féraud, nous conduisons actuellement une mission de contrôle sur l'immobilier du ministère des affaires étrangères. Beaucoup reste à faire, notamment pour déterminer une stratégie de financement pérenne. Nous rendrons nos conclusions début 2023, après avoir effectué une visite à Madrid, où nous observerons les mesures prises dans un pays où les choses sont, de l'avis de tous, bien faites. Je

À titre d'exemple, les crédits de la communication augmentent de 2,5 millions d'euros pour financer la lutte contre la désinformation. Certes, le sujet est important et la somme n'est pas énorme. Mais nous aurions pu la trouver ailleurs, afin d'éviter cette augmentation. De la même manière, 5,4 millions d'euros ont été ajoutés pour financer l'exposition universelle d'Osaka, alors que d'autres lignes budgétaires auraient pu servir. Par ailleurs, le relâchement sur les dépenses de personnel, que j'ai déjà évoqué, me semble plus que critiquable. Enfin, et j'ai eu l'occasion de le dire en commission des finances, je doute très sincèrement de la crédibilité de la trajectoire de la programmation. Lors de nos travaux préparatoires, nos interlocuteurs au ministère semblaient découvrir la programmation des finances publiques sur les trois prochaines années. Or le projet de loi de programmation prévoit au moins 100 millions d'euros d'économies d'ici à 2025 en euros constants. Personne ne semble en mesure d'expliquer comment ce résultat sera atteint, ce qui est particulièrement préoccupant.

Je veux remercier spécial. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, après mon collègue rapporteur spécial Vincent Delahaye, j'évoquerai plus particulièrement

transférée au ministère de l'économie et des finances et Atout France ne fait désormais plus partie des opérations relevant de la diplomatie culturelle et d'influence. Pour ce qui concerne les instituts français à l'étranger, je constate que les moyens sont stables en valeur. Mais cela représente une source d'inquiétude, puisqu'une perte de ressources en volume est à prévoir en raison de l'inflation, souvent un peu plus élevée dans les pays concernés qu'en France, d'autant que ces instituts présentent un un déficit d'environ 43 millions d'euros en 2022 ; celui-ci devrait donc s'accentuer. En effet, les documents budgétaires montrent que certaines dépenses, liées notamment aux salaires, augmentent de manière significative. nous interrogeons donc sur la capacité de la dotation en euros à préserver un niveau d'activité correcte, alors même qu'elle reste stable en valeur. Des amendements ont été déposés en ce sens par certains de nos collègues, et je pense que le Gouvernement devra prendre le temps d'expliquer son intention s'agissant des instituts français et de leur stabilité financière. En matière d'attractivité universitaire, les crédits dédiés au financement des bourses pour les étudiants et chercheurs étrangers s'élèvent à 59 millions d'euros, comme en 2022. Cependant, ce montant stable ne doit pas cacher que ces crédits sont sous-consommés,

Enfin, les crédits du réseau consulaire, hors bourses aux élèves de l'AEFE, s'élèvent à 285,9 millions d'euros et connaissent une hausse de 2 %, bien qu'aucun crédit ne soit dédié l'an prochain à l'organisation d'élections.

a supporté pendant des années la plus grande part des efforts de maîtrise des effectifs de la mission, qui ont entraîné la suppression de 169 ETP entre 2018 et 2021. Cette baisse s'étant révélée difficilement soutenable, le ministère a ainsi recréé 136 ETP et lancé le service France Consulaire, pour mutualiser la prise en charge des appels aux postes consulaires sur le site du Quai d'Orsay situé à La Courneuve. Ainsi, une grande part des efforts réalisés dans le cadre d'Action publique 2022 pour diminuer le nombre d'emplois d'agents publics à l'étranger ont été annulés. On peut bien qu'il est dommage d'annuler si brutalement un effort considérable de réduction d'effectifs ou conclure, comme je le fais, que ces efforts étaient si déraisonnables que le Gouvernement a dû revenir dessus. En tout état de cause, cette situation interroge sur la cohérence de la politique gouvernementale de maîtrise des dépenses publiques. Les moyens de l'AEFE

Par ailleurs, si les crédits pour les bourses aux élèves de l'AEFE augmentent de 10 millions d'euros, nous ne devons pas oublier qu'il faudra faire face, dans le courant de l'année 2023, à la très forte inflation touchant les frais de scolarité dans certains pays du monde. L'impact de ces hausses sur les bourses n'a pas été inscrit dans le budget, et il y a là une vraie source de préoccupation. Car si le surplus nécessaire pour le versement des bourses aux élèves a été pris en charge ces dernières années par la soulte de l'AEFE, la réserve n'est plus aujourd'hui que de 15,5 millions d'euros et devrait être épuisée à la fin de 2023. Ainsi, la question de l'augmentation de ces crédits se posera donc en 2024 ou peut-être même avant. Pour conclure, je souhaiterais rappeler qu'il nous faut considérer cette mission avec attention, parce qu'elle est certainement la seule à subir à la fois les effets de l'inflation et du risque de change. À court terme, les crédits, qui restent À court terme, les crédits, qui restent contraints, demeurent stables en valeur et diminuent très peu en volume. À moyen terme cependant, une baisse en volume de l'ordre de 100 millions d'euros est prévue d'ici à 2025 sur l'ensemble de la mission, comme l'a rappelé mon collègue Vincent Delahaye. Je ne suis pas sûr que cette baisse soit crédible, et je ne pense pas qu'elle soit souhaitable. En effet, les économies antérieures ont mis en tension le réseau et il apparaît désormais nécessaire de redonner les crédits et les effectifs suffisants

nous nous félicitons que les crédits annulés au mois de mars aient bien été rouverts au mois d'août, suivant les recommandations de notre commission. De même, la couverture de 90 % du risque de change des contributions internationales et des opérations de maintien de la paix de mai 2022 est de bonne gestion. Il faudra poursuivre ces efforts en 2023. Ainsi, 27,9 millions d'euros sont prévus pour couvrir le risque change-prix. Mais la hausse des dépenses d'énergie et des dépenses courantes nous fait craindre que les provisions ne soient pas suffisantes. Nous devrons y être attentifs. La politique immobilière à l'étranger reste à réinventer en urgence. Faire dépendre l'entretien normal des bâtiments des recettes exceptionnelles de cessions d'immeubles et du programme 723 du compte d'affectation spéciale était une erreur. En effet, le fonctionnement du le fonctionnement du compte d'affectation spéciale n'a pas permis la mise à disposition de la dotation exceptionnelle de 36 millions d'euros prévue en 2022. Nous serons attentifs à son versement en 2023. Le financement par cessions appauvrit l'État, qui s'essouffle : les ventes deviennent difficiles à réaliser et leur produit est fléché vers le financement des travaux du Quai d'Orsay, à hauteur de 60,8 millions d'euros.

millions d'euros en autorisations d'engagement, afin de permettre la réalisation des schémas pluriannuels de stratégie immobilière. Enfin, nous avons un dernier point d'attention, qui concerne l'application de la réforme de l'encadrement supérieur de l'État au ministère des affaires étrangères. La commission recommandait, notamment, de reprendre le dialogue avec les personnels et d'associer le Parlement à la réflexion. Satisfaction nous a été donnée avec le lancement des États généraux de la diplomatie, qui doivent aboutir au plus tard à la fin du premier trimestre 2023. Nous veillerons au renforcement de notre appareil diplomatique, essentiel dans un monde plus dangereux, instable et de moins en moins prévisible. Je salue les efforts déployés par tous les personnels du ministère pour faire face à ces chocs et crises stratégiques majeures et garantir le rayonnement de la France. La commission des affaires étrangères a donc

par des évolutions réclamées par notre commission, notamment la poursuite de l'augmentation des contributions volontaires aux organisations internationales. Le pilotage du programme est contraint par le poids du réseau et des contributions internationales, qui représentent près de 70 % des crédits. Dans ce contexte, un effort particulier est mené depuis 2017 pour retrouver des marges de manoeuvre et restaurer l'influence de la France. En 2020, aux Nations unies, la France est devenue le sixième contributeur obligatoire, en raison de la baisse de la quote-part française au budget des opérations de maintien de la paix et au budget régulier de l'ONU. Malgré les efforts notables de ces trois dernières années, nous ne sommes que le neuvième contributeur volontaire. L'Allemagne et le Royaume-Uni ont versé respectivement dix fois et cinq fois plus de contributions volontaires que la France en 2020. Pour trouver la réponse adéquate à cette situation, dès 2017, le MEAE s'est doté d'un comité de pilotage des contributions internationales et opérations de maintien de la paix. Celui-ci définit et programme nos contributions volontaires à verser dans l'année. Pour 2023, elles atteindront 58,3 millions d'euros et placeront la France au septième rang des contributeurs globaux. La France a ainsi regagné trois places par rapport à 2019. Outre ce classement amélioré, des résultats concrets sont à mettre à l'actif du ministère. Nous pouvons ainsi nous réjouir d'avoir gardé la tête du département des opérations de paix de l'ONU, d'avoir pesé sur le lancement d'une enquête sur la situation en Ukraine par le bureau du procureur de la Cour pénale internationale ou encore d'avoir intégré le groupe des douze plus grands contributeurs au Fonds de consolidation pour la paix, ce qui nous donne voix délibérative sur la définition des orientations stratégiques. Nous pouvons ainsi orienter l'action du Fonds vers des zones que nous jugeons prioritaires, comme les Balkans ou l'Ukraine. Nous avons aussi été à l'initiative du lancement de la stratégie des Nations unies sur la lutte contre la désinformation, grâce à notre position de premier contributeur aux actions du département des opérations de paix. En matière de sécurité, notre soutien accru à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a constitué un complément utile aux efforts menés sur le dossier du nucléaire Nos contributions volontaires à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) ont permis de soutenir le travail de terrain, tant sur le dossier chimique syrien, que, plus récemment, en Ukraine. La commission des affaires étrangères s'est donc prononcée favorablement

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, il est désormais admis que les luttes d'influence sont au coeur de la compétition mondiale. En la matière, la France dispose d'incontestables atouts : premier réseau culturel au monde, premier réseau éducatif, troisième réseau diplomatique. Pour autant, la place de la France n'est pas immuable. Au cours du précédent quinquennat, le Gouvernement a affiché des ambitions élevées pour la diplomatie culturelle et d'influence de notre pays, ambitions reprises dans une « feuille de route de l'influence » présentée au mois de décembre 2021 par Jean-Yves Le Drian. Pour autant, force est de constater que le fossé s'est creusé entre les discours et les actes. Ainsi, en 2023, les crédits du programme 185 progresseront de 40 millions d'euros à périmètre constant, dont 30 millions iront à l'AEFE. Ce qui nous est présenté comme une hausse Ce qui nous est présenté comme une hausse importante des moyens de l'agence ne vise en réalité qu'à compenser des dépenses supplémentaires : l'aide nécessaire au réseau de l'enseignement français au Liban, l'augmentation, tout aussi nécessaire, du point d'indice et la mise en place d'un nouveau statut pour les pour les personnels détachés. Sur ce dernier point, les crédits ouverts par le projet de loi de finances ne permettront de couvrir que la moitié du surcoût. lors de votre audition devant notre commission, vous vous êtes voulue rassurante, en nous indiquant que l'autre moitié de ce surcoût serait financée par un reliquat de crédits ouverts en 2020. Il n'en est pourtant rien ! Loin d'une augmentation de ses moyens, l'Agence devra donc faire face à une dépense supplémentaire de 7 millions d'euros en 2023. Et cette dépense a vocation à croître dès 2024. Cette stagnation, voire cette régression des moyens de l'AEFE n'a néanmoins pas conduit le Gouvernement à interroger l'objectif présidentiel de doubler les effectifs d'élèves du réseau de l'AEFE d'ici à 2030, objectif qui apparaît désormais

En tout état de cause, l'augmentation du nombre d'élèves ne saurait constituer l'unique boussole de l'enseignement français à l'étranger. En effet, nous avons été alertés sur le risque de développement d'une concurrence entre établissements. C'est pourquoi nous appelons à la mise en place d'une véritable « carte scolaire » établie par l'AEFE, afin de garantir un développement harmonieux du réseau. Par ailleurs, la croissance du réseau ne doit pas être entravée par la question du financement des investissements immobiliers des établissements en gestion directe, qui n'est toujours pas résolue. C'est pourquoi nous proposons qu'une subvention pour charges d'investissement soit inscrite dès le PLF pour 2024. En conclusion, mes chers collègues, vous l'aurez compris, ce PLF ne nous semble pas à la hauteur d'une politique d'influence réellement ambitieuse.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, s'agissant de l'attractivité de la France en matière de mobilité étudiante, la subvention versée à Campus France sera stable.

notre pays est en perte de vitesse dans ce domaine. Ainsi, entre 2014 et 2019, la France est passée de la quatrième place à la septième place dans le classement des pays accueillant le plus d'étudiants en mobilité.

et aux bourses étudiantes, qui stagnent, et les ambitions affichées. Je rappelle que le budget allemand consacré aux mobilités entrantes est trois fois supérieur au nôtre. la durée moyenne des bourses doit être allongée. Actuellement, celle-ci est de moins de six mois, ce qui conduit à un saupoudrage des moyens et ne permet pas de créer un lien pérenne avec les étudiants accueillis. Troisièmement, notre système universitaire souffre- nous le savons depuis longtemps -de son manque de lisibilité, du fait de la coexistence d'écoles et d'universités.

Tout au plus savons-nous que 2 millions d'euros leur seront consacrés en 2023. Elles seront en outre financées par des économies dites de « constatation ». Je ne sais toujours pas ce que signifie « économies de constatation J'espère qu'on pourra me l'expliquer un jour ! Enfin, les moyens dévolus au réseau culturel, instituts français et alliances françaises, seront également stables l'année prochaine. Cette stabilité interroge, dans un contexte de fragilisation de certains établissements du fait de la crise sanitaire et de l'inflation qui touche de nombreux pays.

mon collègue Guillaume Gontard et moi-même avons rapporté pour avis les crédits du programme 151 pour la commission des affaires étrangères et de la défense. Lors de sa réunion du 16 novembre, la commission a émis un avis positif sur l'adoption de ces crédits. Le programme 151 comporte, comme chaque année, les ressources dédiées aux Français à l'étranger et aux affaires consulaires. Elles se répartissent entre trois grands postes de dépense : le service public pour nos compatriotes à l'étranger pour environ 60 % des crédits

L'année 2023 marquera par ailleurs une forme de « retour à la normale » pour le programme 151, du fait de l'absence d'élection directe à l'échelle nationale. Pour mémoire, l'organisation des élections présidentielles, puis législatives qui se sont tenues cette année avait donné lieu à un abondement spécifique de 14 millions d'euros en loi de finances pour 2022. Nous relevons toutefois que, pour faire face à cette échéance, le ministère avait réduit ponctuellement sa dotation de financement des bourses scolaires de près de 10 millions d'euros, en s'appuyant sur la soulte de l'agence pour maintenir constant le soutien financier aux familles expatriées. Ces deux opérations budgétaires s'étant en quelque sorte « mutuellement neutralisées » en 2022, c'est bien une stabilisation des crédits que nous constatons pour l'année 2023, avec une hausse globale de 5 %. Par ailleurs, nous nous sommes intéressés plus particulièrement au déploiement du service France Consulaire. Ce service est une innovation, qui a été mise en place par le Quai d'Orsay à partir du 13 octobre 2021. Il s'agit d'une plateforme de réponse dématérialisée, qui peut être sollicitée par téléphone ou par courriel par les Français résidant à l'étranger ou de passage à l'étranger. Sur son déploiement, nous retenons deux principaux points de vigilance. Le premier concerne le fait que le service France Consulaire ne saurait servir de prétexte à de nouvelles réductions d'effectifs. Le second a trait au calendrier de déploiement du dispositif, qui est moins ambitieux que les objectifs initialement annoncés. Cette dernière constatation ne remet pas en cause la réussite de l'expérimentation. Elle justifie néanmoins que nous soyons particulièrement attentifs à ce que le déploiement de France Consulaire soit accompagné des moyens adéquats. La parole

de l'étranger, les crédits du programme 151 finançant notamment les bourses scolaires du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, l'AEFE. Les dépenses sociales gérées par les postes consulaires ont connu plusieurs années exceptionnelles du fait de la création en avril 2020 du secours occasionnel de solidarité,

pendant l'ensemble de l'année 2021 s'est traduite par un montant exceptionnel d'aides sociales versées pendant cet exercice : 27 millions d'euros, dont 12 millions pour le seul versement des aides SOS covid. À cet égard, l'augmentation d'environ 1 million d'euros de l'enveloppe de financement des aides sociales en 2023 ne saurait sérieusement être présentée comme une compensation à due concurrence de la suppression du dispositif SOS covid, dont le montant atteignait plus de 10 millions d'euros en année pleine. Cette augmentation limitée du budget de financement des aides sociales consulaires est d'autant plus préoccupante que de nombreux facteurs sont susceptibles de faire croître le nombre de nos compatriotes en situation précaire au cours de l'exercice 2023. Face à une inflation qui devrait atteindre plus de 6 % à l'échelle mondiale en 2023, les aides sociales qui ne seront pas revalorisées risquent de voir leur valeur réelle diminuer. Enfin, cette dégradation de la situation économique intervient alors que l'administration consulaire nous a indiqué qu'elle ne disposait pas d'un instrument de mesure du taux de non-recours à ces aides ; celui reste donc inconnu. Sur le sujet des bourses scolaires, je rappelle que les bourses distribuées par le réseau de l'AEFE sont financées par une enveloppe spécifique prélevée sur les crédits du programme 151. En 2021, ces bourses ont profité à plus de 24 000 élèves répartis dans 137 pays différents, pour un coût total de 103 millions d'euros. Toutefois, mes chers collègues, j'attire votre attention sur les défauts de budgétisation de l'enveloppe de financement des bourses scolaires. Dans les dernières années, et en particulier en 2022, les crédits inscrits en loi de finances initiale ont été inférieurs au coût réel du financement des bourses scolaires. Cette différence était rendue possible par l'existence d'un excédent de trésorerie de l'Agence, appelé « soulte qui a financé pendant plusieurs exercices successifs le solde entre les crédits votés en loi de finances et le coût réel des bourses. Ce mécanisme nuit à la clarté et à la lisibilité du dispositif de financement des bourses scolaires et nous serons attentifs à ce qu'à l'avenir les crédits votés annuellement se rapprochent du coût réel des bourses scolaires. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je partage avec mes collègues rapporteurs spéciaux la satisfaction de voir progresser les crédits accordés à la mission « Action extérieure de l'État », et plus particulièrement ceux qui sont consacrés à la diplomatie culturelle et d'influence. Dans le contexte très préoccupant que nous connaissons, cette évolution mérite d'être saluée.

Faut-il rappeler que le rythme annuel moyen de la croissance des effectifs est très en deçà de celui qui serait nécessaire pour atteindre l'objectif présidentiel d'un doublement des effectifs d'ici à 2030 ? Pour la première fois, madame la ministre, je constate que vos services reconnaissent un certain décalage entre l'ambition affichée et la réalité de la mise en oeuvre ... Dès 2018, notre commission avait, pour sa part, émis de sérieux doutes sur la faisabilité L'un des principaux défis structurels posés par la croissance du réseau est celui de l'entretien et de l'agrandissement des établissements en gestion directe. Or l'AEFE n'a plus l'autorisation d'emprunter pour effectuer des travaux, quand les établissements conventionnés et partenaires, eux, peuvent recourir à la garantie de l'État. L'opérateur est dans une impasse financière, alors que les besoins de financement immobilier sont évalués à 300 millions d'euros sur les cinq prochaines années. C'est pourquoi, sur ma proposition, la commission a adopté un amendement visant à autoriser de nouveau l'AEFE à emprunter. Celui-ci ayant été déclaré irrecevable, il ne sera pas discuté en séance ; je souhaite néanmoins, madame la ministre, connaître votre position sur ce sujet. J'ajoute que la commission de la culture a également décidé de proposer la suppression de l'article 41 Mon deuxième bémol porte sur les instituts français et les alliances françaises. La stabilisation de leur budget risque de se heurter, dès les premiers mois de l'année 2023, à la dégradation de leur situation financière compte tenu de l'effet ciseaux provoqué par l'inflation. Des redéploiements de crédits vers les structures les plus fragilisées devront sans doute être envisagés. Mon troisième et dernier point de vigilance a trait à l'Institut français de Paris, dont le modèle économique est en pleine évolution.

Je déplore d'ores et déjà qu'un volet « moyens » ne soit pas à l'ordre du jour de ce nouveau COP. Madame la ministre, quelles sont vos intentions en la matière ? Sous le bénéfice de ces observations, la commission de la culture a émis un avis favorable sur l'adoption des crédits du programme 185. Mes chers

on parle d'une centaine de nouveaux postes. C'est bien ! Mais ce ministère est certainement celui qui a le plus souffert, depuis dix ans, des cures d'austérité : plus du tiers de ses effectifs ont été perdus.

dix ou vingt fois plus de personnel pour soulager nos équipes consulaires, qui ont été en première ligne lors de la crise du covid-19 et dont nous continuons d'avoir besoin ! J'ai la chance de représenter au Sénat les Françaises et les Français qui vivent hors de France. Je suis témoin tous les jours-

la mesure de l'urgence écologique. Celle-ci devrait pourtant être l'une des principales préoccupations s'agissant de déterminer et de financer les actions de l'État, y compris à l'étranger. Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste -Solidarité et Territoires ne votera pas les crédits de la mission budgétaire « Action extérieure de l'État ». La parole

Ce budget est au service d'un objectif primordial, qu'a rappelé le Président de la République lors de la dernière conférence des ambassadeurs, en septembre : faire en sorte que la France demeure « une puissance d'équilibres capable par ricochet d'appuyer l'autonomie stratégique de l'Europe, capable aussi d'agir efficacement en faveur du multilatéralisme et de trouver des voies diplomatiques de résolution des conflits. vient avant tout muscler notre action diplomatique en Europe et dans le monde, face aux nombreux défis qui nous préoccupent. Comme vient de l'expliquer notre collègue rapporteur pour avis André Gattolin, la poursuite de la hausse de nos contributions volontaires aux organisations internationales y participera pleinement. Je m'en réjouis, car les efforts de ces dernières années produisent des résultats tangibles, aussi bien dans le domaine du maintien de la paix qu'en matière de sécurité internationale.

Ce souffle nouveau ne sera pas de trop, face à la multiplication des crises internationales. C'est dans ce contexte que le budget du centre de crise et de soutien sera lui aussi rehaussé de 600 millions d'euros en 2023. efforts, auprès de nos postes diplomatiques, pour venir en aide à nos compatriotes en danger dans les zones de conflit. Je les salue ! J'aimerais d'ailleurs soulever un enjeu qui me paraît crucial et urgent : celui du renforcement

Nous resterons très vigilants, par ailleurs, quant à la sécurisation de nos emprises diplomatiques et consulaires, en particulier lorsqu'elles se situent dans des zones instables et sujettes à des risques d'attentat.

à la promotion de l'influence culturelle et interculturelle française à l'étranger, au niveau de diffusion de la langue française et au développement de l'enseignement francophone. À cet égard, je me félicite

Je veux remercier nos agents qui sont au contact de nos concitoyens, établis hors de France ou seulement de passage ; ils les protègent et les accompagnent dans diverses situations de détresse. Ces dernières années, plusieurs pays ont pris la décision de réduire la couverture de leurs réseaux consulaires dans le monde. Tel n'est pas le chemin qu'a emprunté la France. Mieux encore, nous avons choisi de lancer un vaste chantier de modernisation

a ainsi été proposée pour qu'ils puissent faire face, comme leurs concitoyens en France, à cette situation unique. Je me félicite que cette aide ait d'ailleurs été reconduite en 2021 puis en 2022, tant elle était nécessaire.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la France a fait le choix d'un modèle que de nombreux pays nous envient et tentent d'imiter : celui d'un réseau complet, à la fois diplomatique, consulaire, éducatif, culturel et économique. C'est un héritage exceptionnel, que nous avons le devoir de préserver. Madame la ministre, vous allez nous inviter à nous réjouir de l'augmentation des crédits et du nombre de postes. Il est vrai que cette inversion de la courbe budgétaire, que nous appelons de nos voeux depuis longtemps, est bienvenue. l'augmentation de 5 % des crédits de la mission « Action extérieure de l'État » n'est malheureusement ni structurante pour l'avenir du ministère ni l'expression d'une volonté politique de changement, puisqu'elle sera en grande partie absorbée par l'inflation et par la dépréciation de l'euro. Par ailleurs, le saupoudrage des crédits ne permettra de financer aucune aucune nouvelle mesure. La création de 106 ETP, présentée comme le « réarmement » de la diplomatie française, est loin de compenser la suppression de 160 postes sur la seule année 2019. L'« équipe France » que forment l'ensemble des personnels et nos conseillers des Français de l'étranger a fait preuve d'une grande résilience durant la pandémie et d'un élan spontané de solidarité à chaque crise, empêchant le tissu social de se déchirer. S'ils méritent notre reconnaissance, ils ont surtout besoin que les moyens humains et financiers qui leur sont alloués soient J'en viens maintenant à notre action consulaire, en particulier à la qualité des services publics offerts aux Français de l'étranger et à notre politique des visas. Les consulats devraient être les premiers lieux d'accueil de nos compatriotes à l'étranger, mais ils sont de moins en moins accessibles. Paradoxalement, les usagers parviennent très difficilement à obtenir un rendez-vous, faute de personnel. Quant à la dématérialisation, censée faciliter leurs démarches les plus élémentaires, elle prive une partie de la population d'accès aux services publics. Elle doit vraiment demeurer un outil additionnel, par ailleurs très utile, au lieu d'être utilisée comme le revers d'une politique de suppression de postes et d'économies. Le choix de l'externalisation montre lui aussi ses limites : le service France Consulaire, mis en place pour pallier la suppression des accueils téléphoniques dans les consulats, nécessite en définitive des crédits importants, de l'ordre de 1,9 million d'euros en 2023, et mobilise de surcroît des personnels du ministère à Paris. Est-il vraiment judicieux de continuer à supprimer des emplois dans les consulats pour les déployer ensuite à Paris ou à Nantes ?

La création de 18 ETP au sein du réseau consulaire, dont 7 en administration centrale et 11 à l'étranger, est de toute évidence très insuffisante. L'augmentation des délais de prise de rendez-vous a engendré la création de plateformes privées censées pallier les carences de l'État ou, pire, l'apparition de trafics illégaux de vente de rendez-vous

certaine rancoeur envers notre pays, pareils refus étant souvent vécus comme des humiliations. À l'instar de cette politique qui ternit l'image de notre pays à l'étranger, la réforme de la haute fonction publique abîme notre diplomatie professionnelle à l'heure où les grands bouleversements géopolitiques requièrent la plus grande expertise. Après avoir imposé cette réforme sans concertation, pourquoi ne pas utiliser les États généraux de la diplomatie pour présenter un projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Europe et des affaires étrangères ? J'aimerais maintenant évoquer le deuxième pilier de notre présence à l'étranger : notre réseau éducatif et culturel. En 2018, le Président de la République demandait à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger de doubler le nombre d'élèves en un temps record,

qui portent en eux la philosophie de l'école publique française, dont la mission est de défendre nos valeurs l'enseignement de notre langue. Les 30 millions d'euros supplémentaires prévus pour l'Agence en 2023 ne compenseront pas l'annulation de crédits de 33 millions d'euros subie en 2017.

principalement gérés par la Mission laïque française. Que reste-t-il alors pour les rémunérations de nos personnels, dont le pouvoir d'achat est amputé par l'inflation et par des taux de change très défavorables dans certains pays ? de nos établissements, qui accumulent les difficultés ?

La dotation allouée aux bourses scolaires est en hausse de 11 %, mais elle revient en réalité à son niveau de 2021. La conjugaison de la croissance du nombre d'élèves et de la crise économique prolongée engendre, de fait, une augmentation des demandes de bourses dans nos établissements. Nous plaidons donc pour que l'enveloppe soit revue à la hausse afin d'assurer la mixité sociale, préserver l'attractivité de notre réseau et de répondre à tous les besoins. Il en va de même pour nos établissements culturels, dont les ressources propres ont été réduites par les confinements. Leur stabilisation budgétaire témoigne d'un manque d'ambition pour notre diplomatie culturelle. Comment atteindre l'objectif fixé par le chef de l'État, celui d'ouvrir dix nouvelles alliances françaises chaque année, sans moyens supplémentaires ? Nos instituts français auraient eux aussi mérité un soutien, alors qu'ils continuent de souffrir sur le terrain. D'une part, s'ils ont su se moderniser grâce à l'ouverture de cours en ligne, ils sont aujourd'hui fortement concurrencés par d'autres organismes. D'autre part, la suppression des postes des directeurs des instituts français de Fès, de Tanger et d'Agadir oblige nos consuls généraux à exercer à plein temps deux métiers différents

nous ne pouvons que regretter que notre audiovisuel extérieur ne soit pas plus soutenu face à une concurrence internationale accrue. Enfin, notre développement économique s'appuie sur un réseau formidable d'acteurs. Notre « équipe France », composée d'Atout France, des conseillers du commerce extérieur, de la Chambre de commerce internationale et de Business France, ne doit pas être oubliée. En effet, nos entrepreneurs français sont des soutiens pour les exportations françaises vers leur pays de résidence, et beaucoup d'artisans développent localement les savoir-faire français, ce qui renforce l'image déjà plutôt positive dont bénéficie notre pays. Comme dans bien d'autres domaines, nous possédons les acteurs et les outils ; sans hésiter, donnons-leur les moyens d'être à la hauteur de notre ambition collective

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, en cette période de résurgence des conflits sur le continent européen et d'aggravation des crises de tous ordres au niveau mondial, la France se doit de disposer d'une action extérieure forte, d'un programme ambitieux de solidarité internationale et d'un réseau diplomatique à la hauteur de ces ambitions. Nous accueillons favorablement l'augmentation des crédits alloués à la mission « Action extérieure de l'État », ainsi que le relèvement de 106 ETP du plafond d'emplois du ministère de Mais ces corrections, nous le savons tous, sont loin de réparer les dégâts subis sur une longue période par nos moyens d'action extérieure. De surcroît, à l'insuffisance des moyens s'ajoute la rupture de confiance qu'a provoquée l'entêtement du Gouvernement à mettre en cause envers y compris le Sénat -le modèle de recrutement et le statut de notre corps diplomatique. Là encore, les corrections apportées n'effacent pas tout. Le Quai d'Orsay a connu, au mois de juin, une grève sans précédent, qui laisse des traces,

Le risque de fragilisation de la qualité de notre diplomatie reste réel, alors même que son excellence est largement saluée. Au-delà de ces remarques budgétaires, je veux consacrer les quelques minutes qui me sont imparties à souligner le caractère stratégique de notre engagement diplomatique dans la prévention des conflits. Il s'agit de bien plus, en effet, que d'une question budgétaire. Nous ne saurions nous contenter de préparer la guerre. Dans ce monde plein de convulsions, nous devons mettre au coeur de nos priorités la prévention de celle-ci et la recherche en toutes circonstances d'une solution- diplomatique, politique, économique -aux conflits qui menacent.

Face à une mondialisation hyperconcurrentielle, qui mine les solidarités et fait naître des insécurités globales, alimentaires, sanitaires, migratoires, sociales, énergétiques,

de notre stratégie de promotion d'une paix mondiale globale. Je prendrai quelques exemples d'actualité. Premier exemple : la guerre en Ukraine. Je ne reviendrai pas sur les sous-estimations, l'aveuglement et les échecs successifs qui ont conduit à négliger les accords de Minsk-

Il y a 10 000 formules différentes : des régions plus décentralisées comme prévu par les accords de Minsk, avec reconnaissance, par exemple, de la co-officialité de la langue russe, des territoires sous protection internationale, des formules d'autodétermination ... » Comment être utile

Faisons-nous des COP un objectif de sécurité stratégique ? Le cas échéant, de quels moyens diplomatiques supplémentaires nous dotons-nous pour ne pas aller, de COP en COP, d'échec en échec ? Troisième exemple : l'échec de Barkhane. Quelles conclusions en tirons-nous, au-delà des seuls aspects militaires ? En effet, l'échec est avant tout politique et géostratégique. Qui redéfinira nos relations avec les pays du Sahel autrement qu'en s'enfonçant dans les ruptures actuelles,

en matière de sécurité collective sans de puissants efforts politiques et diplomatiques visant à relancer les initiatives internationales de la France dans tous les domaines : pour une solution politique aux conflits, mais, aussi et surtout, pour en éradiquer les racines ; pour un nouvel ordre économique ; pour une transition climatique juste ; pour la sécurité alimentaire ; pour les droits des femmes ; pour le respect d'un droit international qui ne soit plus régi par le « deux poids, deux mesures

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la présidence française de l'Union européenne, au premier semestre, a été une grande réussite, grâce au professionnalisme et à l'engagement de nos diplomates, que je tiens à saluer dès le début de mon propos. La France dispose du troisième réseau diplomatique mondial, mais celui-ci avait perdu 50 % de ses effectifs en trente ans. Jean-Yves Le Drian a donc eu raison de mettre un coup d'arrêt à la baisse continue des moyens du Quai d'Orsay.

la réforme de la haute fonction publique au corps diplomatique a incité le Président de la République à organiser des États généraux de la diplomatie. La semaine dernière, notre commission a rencontré l'ambassadeur Jérôme Bonnafont, rapporteur général des États généraux, et son équipe, qui nous ont la modernisation des ressources humaines du Quai d'Orsay constitue le grand enjeu de cette réflexion. L'évolution des missions et des métiers diplomatiques et consulaires envisagée me paraît encourageante. et d'influence », je répondrai aux détracteurs de l'ambition présidentielle de doubler la taille du réseau de l'enseignement français à l'étranger d'ici à 2030. En 1990, lors de la création de l'AEFE, le réseau comptait 499 écoles. ans plus tard, il n'en comptait plus que 470. Lorsqu'Emmanuel Macron a partagé sa volonté de développer le réseau en 2018, l'AEFE n'était toujours pas parvenue à recouvrer le nombre d'écoles Le nouvel élan porté par le Gouvernement a permis de passer de 495 à 560 écoles françaises à l'étranger en quatre ans ; c'est historique.

l'AEFE est confrontée à un conflit d'intérêts : il lui est demandé de développer un réseau destiné à faire concurrence aux 68 établissements qu'elle administre en gestion directe.

Les 498 écoles privées mériteraient d'ailleurs d'être auditionnées par les rapporteurs du programme 185. En effet, qui n'entend qu'une cloche

je rends hommage à nos élus des Français de l'étranger engagés en matière de solidarité, ainsi qu'à la Fédération internationale des accueils français et francophones d'expatriés, la Fiafe, qui a été reconnue d'utilité publique le mois dernier.

et dans le monde », qui regroupe les moyens de l'action diplomatique de la France, j'ai pu constater les effets positifs de la hausse des contributions volontaires de la France aux organisations internationales lors de la visite de la délégation parlementaire au siège de l'Organisation

la place de la France dans le monde, chère au général de Gaulle, qui se joue là. Peut-être les débats leur rappelleront-ils que l'influence ne se paie pas qu'en mots. Enfin, la Première ministre Élisabeth Borne a appelé les ambassadeurs à renforcer leur relation avec les élus des Français de l'étranger et a fait de la simplification de la vie de nos compatriotes à l'étranger

faire comme si la guerre ne bousculait pas les équilibres européens, que nous espérions stables et consolidés depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette agression doit nous inciter à la prudence, à la modestie et à la vigilance. Après la pandémie, l'agression russe impose une nouvelle fois à l'Union européenne un devoir de solidarité. Il n'est pas question de faire profil bas ou, pire, de baisser la garde- bien au contraire ! Mes chers collègues, nous entendons les réserves émises sur le programme 185. Les conclusions des rapporteurs soulignent que l'augmentation de 13 millions d'euros de l'enveloppe budgétaire consacrée à la diplomatie culturelle et d'influence n'est pas à la hauteur des ambitions affichées par l'exécutif. Sans être adepte du « toujours plus », le groupe RDSE est bien conscient des effets de l'inflation, celle-ci demeurant plus sévère hors de nos frontières que dans l'Hexagone. La compenser intégralement serait une prouesse, puisque cela supposerait une adaptation pays par pays.

de voeux pieux ou d'incantations. Mes chers collègues, le « toujours plus » qui est parfois de mise dans les discussions budgétaires est souvent une façon commode de se donner bonne conscience. De même, la critique, acceptable quand elle est juste et raisonnable, se révèle vaine lorsqu'elle devient systématique. occulte-t-elle souvent les avancées positives que les perspectives budgétaires permettront de concrétiser. Or les lignes tracées pour 2023, sans être flamboyantes, ont l'immense mérite mérite d'être pragmatiques. Ainsi, les deux tiers des 30 millions d'euros supplémentaires octroyés à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger financeront la hausse du point d'indice des enseignants et compenseront en partie la mise en place du nouveau statut de détaché. les 10 millions d'euros dédiés au soutien au réseau d'enseignement du français au Liban sont bien plus qu'un heureux coup de pouce, dans un pays fracturé. Je ne cache pas que je me montrerai plus sévère avec la stratégie Bienvenue en France, destinée à l'accueil des étudiants étrangers. Celle-ci reste bien timide et souffre de la comparaison qui peut être dressée avec les initiatives prises outre-Rhin. Si la France occupait le quatrième rang des pays d'accueil en 2015, elle est désormais septième. Nous consacrons 64 millions d'euros aux bourses étudiantes ; ce budget est trois fois supérieur en Allemagne et s'élève à 266 millions d'euros pour l'Australie.

s'agit sans doute du maillon faible de cette politique, car c'est bien en accueillant et en formant les élites de demain que nous consoliderons notre influence future de manière durable. Notre attractivité ne se résume pas au déroulement d'un tapis rouge pour les entreprises étrangères porteuses de capitaux. Elle passe aussi par un patient et discret travail d'influence, d'accueil et de formation. Je tenais à rappeler ces quelques chiffres avant d'aborder le programme 105, qui est une priorité de la mission « Action extérieure de l'État ». La progression de 6,6 % de ses crédits traduit une volonté politique qu'il nous faut saluer.

Souvenons-nous que les agents animant le troisième réseau diplomatique mondial ont été sur le pont lors de la pandémie, favorisant le rapatriement de plus de 370 000 de nos ressortissants. Ils ont aussi facilité l'évacuation de 3 000 personnes d'Afghanistan, pays plongé dans un obscurantisme accablant. Par ailleurs, nous n'ignorons pas les interrogations liées à la politique immobilière : elles ont fait l'objet de propositions sérieuses de la commission des affaires n'hésitons pas évoquer l'épineuse question de la spécificité des parcours des diplomates, remise en cause par la disparition de l'École nationale d'administration (ENA). Comme vous tous, mes chers collègues, nous avons été sensibles aux inquiétudes provoquées par l'application de la réforme de l'encadrement supérieur de l'État au ministère des affaires étrangères.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, demain, la diplomatie sera plus nécessaire que jamais. Ce constat, nourri par l'inquiétante marche du monde, voilà déjà longtemps que nous le faisons. faisons. L'année écoulée, loin de l'infirmer, aura néanmoins constitué une rupture, un basculement accéléré vers une nouvelle ère. Elle aura fait de notre conviction une évidence. le réveil des ambitions impérialistes est désormais acté, le recours à la force désinhibé, et les cadres internationaux contestés. Une nouvelle géographie des tensions et des rapports de force se dessine, amplifiée par les défis de notre temps, qu'ils soient climatiques, énergétiques, alimentaires ou démographiques. Ce débat a permis de rappeler que c'est précisément quand le monde devient plus instable, plus imprévisible et plus dangereux que la mission de nos diplomates se révèle plus essentielle encore.

Ceux qui relèvent de la mission « Action extérieure de l'État » progresseront de 5,2 % en 2023, s'établissant à 3,2 milliards d'euros. Naturellement, nous nous en réjouissons et vous remercions, madame la ministre, d'avoir obtenu cette avancée inédite. il ne suffit pas d'approuver ces crédits, par ailleurs modestes au regard de ceux qui sont accordés à d'autres ministères. Nous devons surtout nous interroger sur les conséquences, pour notre politique étrangère, de la montée des périls et de l'essoufflement du multilatéralisme. l'agression russe en Ukraine a agi comme le révélateur du nouvel état des relations internationales. Bien sûr, le courage admirable et la détermination de la nation ukrainienne, comme d'ailleurs la contestation populaire en Iran ou en Chine, ébranlent les certitudes de ceux qui annonçaient déjà le triomphe des régimes autoritaires sur les démocraties. Néanmoins, un constat s'impose : les autocrates, quelle que soit leur obédience, ne célèbrent plus seulement la primauté de la force sur le droit, ils la mettent en pratique. Le 24 février fut la violente affirmation de cette tendance de fond, qui nous interroge profondément. Quelles conclusions devons-nous en tirer pour notre pays et pour notre diplomatie ? Les formats doivent-ils être adaptés ? La France a entrepris de concentrer ses personnels vers les zones de croissance en Indo-Pacifique. Doit-elle poursuivre dans cette voie et dans quelles conditions ? Ne doit-elle pas d'abord réexaminer l'état de ses forces en Europe ? En quelques semaines, la guerre en Ukraine a balayé nos vieilles certitudes et mis un coup d'accélérateur aux recompositions géopolitiques qui couvaient. Les exemples ne manquent pas : hier, l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'Otan était inimaginable, elle est aujourd'hui quasiment actée. La Russie s'est profondément et durablement éloignée de l'Europe pour se rapprocher de la Chine. Une Chine qui tire d'ailleurs consciencieusement tous les enseignements de cette guerre impliquant les pays occidentaux, même si ses plans sont également contrariés par les déboires de son partenaire russe, qui s'enferre dans son isolement. Prenons garde toutefois, la condamnation de Moscou n'est pas unanime, tant s'en faut C'est une autre des leçons de la guerre en Ukraine qu'il nous faut regarder en face : le temps où les positions occidentales donnaient le aux relations internationales est révolu. Les positions du G77 expriment la réticence et, parfois, le refus de soutenir les motions occidentales condamnant l'invasion russe. La position de l'Inde, allié stratégique et ami, nous interpelle également. Elle regrette que cette guerre affaiblisse son allié russe en Asie, déplore les retards de livraison d'armement russe, mais tire aussi parti de l'affrontement en achetant en quantité un pétrole russe à prix cassé. Enfin, l'humanité se montre toujours incapable d'apporter une réponse globale au changement climatique- quelle meilleure illustration de l'affaiblissement du multilatéralisme ? Les opinions publiques se mobilisent, les États sont jugés responsables et sont de plus en plus souvent condamnés par la justice ... Et pourtant, la COP27 n'a guère convaincu. le fonds pour les pertes et préjudices reste à construire et, faute d'élan, il a semblé nécessaire d'annoncer un sommet à Paris en 2023, avant la prochaine COP. Madame la ministre, vers quelles perspectives nous ? Dans ces temps troubles, plus que jamais, la France a besoin d'une diplomatie forte. Elle doit tout d'abord pouvoir tenir son rang. Nous sommes un État doté, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, disposant du troisième réseau diplomatique au monde. Membre fondateur de l'Union européenne, la France a un positionnement géographique stratégique, au coeur de l'Europe, qui fait d'elle un trait d'union entre les pays du Nord et le bassin méditerranéen. place nous oblige et nous donne une responsabilité particulière : celle de tenir le positionnement singulier qui a toujours été celui de notre pays. Nous sommes tout à la fois un allié loyal, fiable et efficace au sein de l'Otan, et un promoteur de l'autonomie stratégique européenne. Sachons cultiver cette position équilibrée. La France parle à tout le monde, sans jamais renier ses valeurs- nous en avons fait l'expérience commune aux États-Unis ces derniers jours, madame la ministre. Elle répond au désir de France que les sénateurs constatent dans toutes leurs missions à l'étranger. Face à tous ces enjeux, le PLF pour 2023 amorce la fin de l'éreintement. Mais les temps d'appauvrissement de notre diplomatie ont tant duré que cela ne peut être qu'une première étape. Certes, l'attrition des personnels connaît un réel coup d'arrêt, avec 106 ETP créés. C'est un début, mais c'est encore trop peu, quand on les compare aux 3 000 postes que votre département a perdus depuis 2007. Surtout, on ne sait toujours pas comment ceux-ci seront répartis- vous nous éclairerez sur ce point, madame la ministre. On nous annonce un renforcement des capacités d'analyse politique et des implantations dans l'immense Indo-Pacifique. Ne faudrait-il pas toutefois concentrer ces moyens sur une politique en particulier, pour garantir l'impact de l'effort consenti ? Je pense notamment au renforcement des équipes de nos consulats, qui ont tant souffert des restrictions budgétaires passées. l'oublions pas, s'ils sont le guichet unique pour nos concitoyens vivant hors de France, ils le sont aussi pour les étrangers qui souhaitent s'y rendre. Le traitement des demandes de visas constitue donc la première étape d'une politique migratoire plus efficace. À ce titre, la façon dont on a créé une différence de traitement entre l'Algérie et le Maroc en matière de visas continue de poser des problèmes, même si des évolutions sont en cours. du PLF doit être un moment de clarification pour nos compatriotes : la France a plus que jamais besoin de diplomates et de moyens pour défendre ses intérêts, dans un monde devenu plus dangereux, plus difficile à anticiper et à comprendre- monde sur lequel nos leviers d'action pourraient, si l'on n'y prend pas garde, perdre de leur efficacité. Pour toutes ces raisons, le Sénat attend des États généraux de la diplomatie qu'ils confortent le corps diplomatique, lui qui a été si meurtri par la réforme qui le vise et auquel nous rendons régulièrement un hommage appuyé. ne serait-ce que pour son action en faveur du rapatriement de nos compatriotes pendant la pandémie, l'évacuation de Kaboul, ou la gestion du dossier nucléaire iranien. Cette réforme du corps diplomatique a soulevé beaucoup d'hostilité contre elle,

Si le Parlement avait eu voix au chapitre, peut-être aurions-nous évité la grève des personnels du Quai d'Orsay massivement suivie en juin dernier. Il s'agissait de la première depuis deux décennies- c'est dire le ressentiment de nos diplomates. C'est un signal pour nous tous. Ainsi, il nous faut désormais apaiser ce trouble

Je n'en citerai qu'une, très importante : la consultation des commissions des affaires étrangères du Parlement avant la nomination aux postes d'ambassadeur les plus importants, par exemple dans les grands pays européens, à Pékin, Washington ou au Conseil de sécurité des Nations unies. Il s'agirait en fait d'étendre le dispositif de l'article 13 de la Constitution, qui prévoit déjà la consultation des commissions parlementaires compétentes pour une cinquantaine de postes d'importance dans d'autres domaines- ce serait un signal en manière d'hommage à l'action du Parlement dans ce domaine. En tout état de cause, soyez assurée, madame la ministre, que le Sénat restera vigilant et mobilisé sur ce sujet fondamental pour notre pays. Nous participerons à vos travaux ; nous vous tendons la main pour faire en sorte que l'apaisement suive l'orage.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, après avoir connu une pandémie, le monde connaît à présent de grandes tensions. Le 24 février dernier, la Russie a envahi l'Ukraine, ramenant la guerre sur notre continent. Ce conflit est l'affaire de tous les Européens.

Elle l'a fait lors de la crise sanitaire, en contribuant à la mise en place d'un emprunt commun au sein de l'Union. Ce mécanisme a permis de donner corps à la solidarité européenne et a constitué une véritable avancée. Il y a un pacte vingt fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde », nous disait le général de Gaulle. Notre pays est en effet porteur d'un idéal et de valeurs qui ont, plus d'une fois, influencé le cours de notre histoire la liberté, bien sûr, mais également l'égalité femmes-hommes, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ou encore le destin commun des peuples européens. Il faut préserver la capacité de notre pays à se faire entendre. D'autres pays investissent massivement dans leur diplomatie et se donnent ainsi les moyens de gagner en influence et de peser sur le cours des événements internationaux. La France ne doit pas se laisser distancer. Les crédits que nous examinons contribuent à maintenir notre influence et revêtent donc une importance toute particulière. À cet égard, nous nous réjouissons que les dépenses de personnel de la mission soient en hausse. La hausse des prix globale explique en partie cette augmentation. Le contexte inflationniste n'épargnant pas pas notre pays- ni aucun autre -, il fait progresser le coût des indemnités de résidence à l'étranger. Il ne doit cependant pas masquer le renforcement des effectifs : 106 équivalents temps plein supplémentaires sont prévus pour 2023. Ces personnels permettent à la France de savoir avec précision ce qui se passe à l'étranger, d'analyser, de comprendre, d'anticiper et d'agir en conséquence. Ils contribuent également à faire rayonner notre culture, nos valeurs, nos entreprises. En effet, la France dispose de l'un des réseaux diplomatiques les plus étendus au monde ; c'est un atout qu'il faut préserver. Dans un monde où la désinformation est une arme redoutable en infectant les réseaux sociaux, il est important d'y voir clair par nous-mêmes. La représentation diplomatique est essentielle pour nous assurer d'une évaluation objective des situations à travers le monde. Il nous faudra également continuer d'investir dans le parc immobilier. Le contexte économique pèse sur ces budgets comme sur ceux qui sont consacrés aux personnels : l'inflation érode l'ensemble des crédits. En outre, la remontée du cours du dollar aggrave encore cette situation, en raison de la position dominante de cette monnaie à l'international. Ces augmentations de crédits se justifient amplement : l'influence fait pleinement partie des objectifs stratégiques de la France. Plus que le rayonnement de notre pays, cette capacité doit nous permettre de renforcer notre poids sur la scène internationale. La diplomatie, en temps de crise, et en temps de guerre, peut sembler accessoire à certains ; il n'en est rien. C'est à travers elle que les alliances se nouent et que les rapports de force évoluent, à condition d'y consacrer des moyens suffisants. la Chine ne s'y trompe pas. Elle consacre ainsi plus de 10 milliards de dollars par an au développement de son influence. La France et ses partenaires européens font face à de graves défis militaires, économiques et écologiques. Ces défis nous placent devant une alternative : y répondre collectivement ou bien céder à l'opportunisme de court terme. Aucun État européen ne peut parvenir seul à l'indépendance stratégique. C'est par la coopération et la diplomatie que nous pourrons développer des solutions de long terme conformes à nos intérêts communs. Le budget pour 2023 maintient globalement les fonds consacrés à ces capacités. Même s'il ne les accroît pas autant que nous le souhaiterions, le groupe Les Indépendants votera en faveur des crédits de cette mission. La

M. Pierre-Antoine Levi. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le budget consacré à la diplomatie culturelle et d'influence en 2023 augmente de 40 millions d'euros à périmètre constant, pour un total de 671 millions d'euros. Les moyens de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sont renforcés à hauteur de 30 millions d'euros, tandis que ceux qui sont consacrés au réseau de coopération culturelle sont stables. Comme cela a été rappelé par les orateurs précédents, en mars 2018, le Président de la République fixait pour objectif au réseau d'enseignement du français à l'étranger le doublement de ses effectifs à l'horizon 2030, soit une cible de 700 000 élèves. Cela correspond à une croissance moyenne de l'ordre de 7 % à 8 %. Depuis cette annonce, et malgré la crise sanitaire qui a ralenti le processus de développement, le réseau de l'AEFE a gagné 72 établissements et plus de 30 000 élèves. Le rythme moyen de croissance annuelle des effectifs est toutefois loin d'être assez soutenu pour atteindre l'objectif présidentiel dans le calendrier imparti. Cette ambition présidentielle se heurte notamment à trois enjeux structurels.

bien formés en nombre suffisant, le plan ne pourra pas fonctionner. Le deuxième enjeu est immobilier : pour se développer et faire face à la concurrence internationale, les établissements déjà membres du réseau ont besoin d'améliorer l'état de leur bâti, voire de l'agrandir.

À l'heure de la définition du prochain schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) pour les années 2023 à 2027, l'AEFE évalue le besoin de financement de l'immobilier des EGD à 300 millions d'euros pour les cinq prochaines années. Le troisième enjeu concerne la régulation de la croissance du réseau, afin d'éviter la concurrence déloyale entre établissements anciennement membres et établissements nouvellement homologués. homologués. À ces enjeux structurels s'ajoutent les crises conjoncturelles auxquelles le réseau peut être confronté : l'invasion de l'Ukraine a par exemple touché directement cinq établissements de la région. La crise inflationniste n'épargne aucune zone géographique et suscite de très vives inquiétudes pour 2023. L'envolée des prix des fluides- le chauffage, l'électricité -renchérit directement les coûts de fonctionnement des établissements. Les établissements en gestion directe du réseau ont reçu pour consigne de ne pas répercuter l'entièreté des surcoûts sur les familles et de trouver un équilibre entre hausse des droits d'écolage et économies de dépenses. En 2023, les droits de scolarité devraient augmenter en moyenne de 8 % dans les EGD. Dans certains établissements, la hausse pourrait même atteindre 10 %, voire 12 %, ce qui nourrit de fortes inquiétudes chez les parents d'élèves.

messieurs les rapporteurs, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, permettez-moi tout d'abord de saluer la qualité de vos interventions successives,

Vous le savez, le contexte international n'a pas été aussi critique et dangereux depuis longtemps. Nous vivons en effet dans un monde en voie de fracturation, un monde plus brutal, plus instable, où les menaces globales se renforcent et où les crises se multiplient, comme vous l'avez rappelé, monsieur le président Cambon. De plus, nous voyons que nos intérêts sont souvent contestés, qu'ils soient politiques ou économiques. Nous sommes confrontés à des menaces qui visent nos ressortissants et nos emprises, des menaces qui se déploient aussi dans le champ numérique ou informationnel, où nous sommes la cible d'opérations de propagande Cette tendance à ce qu'on a pu appeler la « brutalisation » du monde ne date certes pas d'hier, mais elle a pris une ampleur nouvelle il y a neuf mois, lorsque la Russie a choisi d'envahir et d'agresser de ramener la guerre sur le continent européen. Du fait de cette agression, des situations de tension deviennent des situations de crises, énergétique ou alimentaire, par exemple,

en crédits de paiement pour l'ensemble des missions, en augmentation de 543 millions d'euros, soit une hausse de 9 % par rapport à la loi de finances initiale pour 2022.

la hausse des moyens humains en 2023, pour la première fois depuis 1993. Cette hausse va nous permettre de disposer de 106 ETP de plus qu'en 2022. Je vous l'avais dit et je vous le confirme, la répartition de ces nouveaux effectifs concernera très majoritairement la mission « Action extérieure de l'État », prioritairement à l'étranger, pour les deux tiers d'entre eux, comme je l'avais annoncé en commission. Grâce aux moyens de la mission « Action extérieure de l'État », nous pourrons maintenir un outil diplomatique universel, capable de se déployer partout dans le monde et d'agir dans la quasi-totalité des organisations internationales et régionales. La France dispose- dois-je le rappeler ? -du troisième réseau diplomatique mondial : celui-ci compte 163 ambassades, 16 représentations permanentes et 90 consulats généraux. Cette universalité nous permet d'être présents partout et nous met en mesure de parler à tout le monde. C'est essentiel pour promouvoir le dialogue politique entre États, construire des partenariats

Notre outil universel est aussi un atout majeur pour bâtir les coalitions d'action dont nous avons besoin pour agir, à l'ONU et dans les organisations internationales. C'est enfin un outil puissant au service de nos ressortissants,

hausse est bien évidemment liée à la création des nouveaux postes à l'étranger dont notre diplomatie a tant besoin, mais beaucoup également à l'inflation mondiale, qui est supérieure à celle que nous connaissons en France en règle générale. Elle est liée, enfin, à la baisse de l'euro. Dans un contexte de persistance et souvent d'aggravation de la menace en Afrique- on l'a encore vu au Burkina Faso -ou encore en Ukraine- tout le pays est frappé par des bombes, aujourd'hui encore -, les moyens nouveaux du programme 105 concerneront d'abord la sécurité. Ils permettront de sécuriser nos ambassades là où nos agents sont le plus exposés à des situations de crise ou d'instabilité. Nous proposons d'y consacrer 5 millions d'euros en autorisations d'engagement et 3 millions d'euros en crédits de paiement. La progression des crédits du programme 105 bénéficiera à une autre priorité : le numérique. Nous continuerons à consentir des investissements soutenus afin d'améliorer l'efficacité de nos outils, de pallier les inégalités de déploiement selon les pays et de renforcer la cybersécurité de notre réseau. Nous souhaitons allouer une enveloppe de 52 millions d'euros à cette priorité, soit une hausse de 4,4 millions d'euros par rapport à l'année dernière. La communication stratégique est un autre enjeu, de plus en plus important alors que nous sommes confrontés à des opérations hostiles de désinformation et de propagande, souvent d'origine russe, mais pas exclusivement, qui visent à attiser les discours antifrançais sur les réseaux sociaux, notamment en Afrique ou en Europe. Afin de mieux lutter contre ces pratiques, nous souhaitons augmenter de 2,5 millions d'euros les moyens de la direction de la communication et de la presse. Dans son discours de Toulon du 9 novembre, le Président de la République déclarait en effet : « l'influence sera désormais une fonction stratégique, dotée de moyens substantiels [ ...] avec, pour sa déclinaison internationale, un rôle central du ministère de l'Europe et des affaires étrangères ».

sénatrices, messieurs les sénateurs, ces priorités s'accompagneront d'une préoccupation constante : aider et protéger les Français de l'étranger, car le Quai d'Orsay est aussi le grand service public des Français à l'étranger. En 2023, notre action consulaire, portée par le programme 151, pourrait être dotée de 141,1 millions d'euros. Alors que nos compatriotes sont confrontés dans de nombreux pays à des contextes économiques dégradés, ils pourront continuer de compter sur une gamme d'aides sociales inégalées chez nos partenaires. Les bourses scolaires, destinées aux enfants français de nos établissements scolaires, retrouveraient leur niveau de 2021, le budget qui y est consacré

Afin de répondre aux besoins accrus de la communauté française à l'étranger, des crédits supplémentaires seront aussi alloués au titre de l'aide sociale 16,2 millions d'euros en 2023, soit 1 million d'euros de plus par rapport à l'année 2022. Toutes ces aides seront distribuées en lien avec les élus consulaires, qui constituent pour nous un précieux relais des besoins des Français de l'étranger

Mélanie Vogel. Il n'est pas besoin de rappeler l'importance considérable de l'éducation pour les générations de demain. Or les Françaises et les Français de l'étranger doivent, eux aussi, pouvoir accéder à un enseignement de qualité à un coût raisonnable. Le problème, c'est que, après correction de l'inflation, le budget alloué

notamment en raison de la politique du chiffre d'Emmanuel Macron, qui veut doubler le nombre de ces derniers, mais, proportionnellement, avec de moins en moins d'enseignants et de personnels pour s'en occuper. Ce désengagement de l'État profite évidemment au secteur privé, on en fait le constat partout au sein de notre réseau. Or il faut donner à l'AEFE les moyens de fonctionner autrement que par des hausses répétées des frais de scolarité, lesquels frappent les Français de l'étranger

sensible pour 2023, en raison à la fois de l'évolution de l'inflation, notamment dans certains pays, et de l'épuisement programmé de la soulte de l'AEFE.

Les Français qui vivent à l'étranger ne parviennent plus à joindre leur consulat par téléphone ; c'est impossible ! Prendre un rendez-vous pour renouveler un passeport ou une carte d'identité prend un temps considérable.

Cet amendement vise donc à augmenter les effectifs du service public consulaire, qui fait face à une hausse du nombre des tâches qui lui sont confiées sans avoir les moyens de les assumer dans de bonnes conditions. met en péril à la fois la santé des agents concernés, qui font pourtant preuve d'un dévouement exceptionnel- la multiplication des cas de burn-out doit nous alerter -et la qualité du service. Les délais de traitement des demandes ont connu une dégradation qui n'est plus soutenable aujourd'hui.

l'amendement n° II-1233. Dans le plan de relance, 4 milliards d'euros sont consacrés à la rénovation énergétique des bâtiments publics implantés sur le territoire national. Le parc immobilier de l'État à l'étranger, lui, n'est pas concerné. Pourtant, lorsque je fais le tour de nos emprises lors de mes déplacements à l'étranger, je constate que certains bâtiments sont de véritables passoires thermiques ou qu'ils ne sont pas adaptés aux aléas du climat. Alors que les coûts de l'énergie augmentent de manière exponentielle dans la majorité des pays, il devient essentiel d'utiliser davantage les énergies renouvelables et d'essayer d'éviter de gaspiller de l'énergie. Il s'agit donc de rénover l'ancien, mais aussi d'inclure les critères énergétiques dans les plans de construction actuels, ce qui, par exemple, n'a pas été le cas pour les nouveaux bâtiments du lycée français de Tunis. Pour faire baisser la facture énergétique et lutter contre le changement climatique, nous ne pouvons pas compter uniquement sur les efforts individuels de nos compatriotes. Nous devons être collectivement responsables et faire les bons choix pour nos équipements. Il y va des conditions de travail de nos personnels et de l'environnement scolaire de nos enfants. Cet amendement vise à consacrer 15 millions d'euros

Nous comprenons bien qu'il s'agit d'un amendement d'appel, et nous en demandons donc le retrait. À défaut, notre avis serait défavorable.

Mais certaines paroles balayent des milliards, balayent l'engagement de dizaines d'agents du Quai d'Orsay, de centaines de Français qui se mobilisent pour l'Ukraine. Lorsque le Président de la République

Actuellement, 7 millions d'euros sont prévus pour compenser la moitié du surcoût lié à la mise en place d'un nouveau statut pour les personnels détachés dans notre réseau scolaire. Madame la ministre, vous avez indiqué que l'autre moitié de ce surcoût serait financée par un reliquat de crédits alloués aux bourses scolaires.

Dans tous les pays du monde, nos compatriotes subissent la crise économique plus ou moins fortement et constatent la baisse de leur pouvoir d'achat. Cette crise n'épargne personne et affecte malheureusement les plus vulnérables. Les élus des Français l'étranger se sont mobilisés dans les conseils consulaires pour demander des augmentations à hauteur du niveau de vie dans les pays de résidence. Ils ont demandé, par exemple, de passer de 310 à 450 euros par mois au Cambodge et de 357 à 557 euros en Argentine. D'autres, à Londres par exemple, ont voté à l'unanimité des motions en conseil consulaire demandant la revalorisation urgente des taux de base. Nous pouvons déjà anticiper que, malgré l'augmentation des crédits prévue en 2023, l'ensemble des besoins ne pourront être satisfaits. Les estimations de tous les acteurs sociaux et des associations d'entraide locale nous démontrent que cette enveloppe est trop limitée. Alors que la situation est critique pour certaines familles, nous ne pourrons pas procéder à des ajustements à la baisse. Où irons-nous chercher les crédits s'ils n'ont pas été fléchés ? Nous avons donc déposé cet amendement, pour être dans l'anticipation et non la réaction, afin de répondre au mieux à la crise économique qui nous frappe et à la paupérisation de nos compatriotes à l'étranger.

J'aimerais vous proposer l'équivalent pour les Françaises et les Français de l'étranger. Cet amendement vise donc à créer un nouveau programme consacré à l'accompagnement et à la prise en charge de la perte d'autonomie des Françaises et des Français de l'étranger, pour un coût de 5 millions d'euros. Certes, de nombreux Français de l'étranger sont affiliés à la Caisse des Français de l'étranger (CFE), mais beaucoup sont encore attachés à la sécurité sociale. Leurs dépenses de santé peuvent ainsi être couvertes, mais pas leur perte d'autonomie.

à M. Yan Chantrel. Cet amendement vise à créer un pass Culture pour les jeunes Français de l'étranger. Contrairement aux collégiens et lycéens de France, les jeunes Français établis hors de France n'ont pas accès au pass Culture. Ce dispositif, depuis 2017, favorise l'accès à la culture afin de renforcer et de diversifier les pratiques culturelles des jeunes tout en révélant la richesse culturelle des territoires. Or, il est essentiel d'entretenir chez les jeunes Français de 15 à 18 ans établis hors de France des liens forts avec la culture française et francophone, à laquelle ils sont, par définition, moins exposés qu'à la culture du pays d'accueil. Le dispositif du pass Culture pour les jeunes Français de l'étranger doit être ciblé vers des acteurs culturels français établis hors de France, qui en seraient partenaires : alliances françaises, instituts français bien sûr, mais aussi librairies françaises, galeries françaises ou cinémas français. La création de ce pass Culture pour les jeunes Français de l'étranger vise donc un double objectif : encourager les pratiques culturelles en autonomie des jeunes Français établis hors de France et promouvoir les acteurs culturels français établis hors de France,

à M. Yan Chantrel. La multiplication des crises internationales, entre l'épidémie de covid-19 et la crise de l'énergie liée à l'invasion de l'Ukraine, a conduit de nombreuses familles à travers le monde à repenser leurs priorités. Cela n'a pas été sans conséquence sur la mobilité internationale des étudiants. L'attractivité des établissements d'enseignement supérieur français est mise à mal, alors qu'elle avait déjà baissé depuis 2019 avec le décuplement des frais universitaires pour les étudiants extracommunautaires. Face à ces difficultés, Campus France a plus que jamais besoin de moyens supplémentaires pour attirer davantage et mieux accueillir les étudiants étrangers dans les établissements d'enseignement supérieur français. C'est pourquoi cet amendement tend à abonder le programme « Diplomatie culturelle et

Elle est garante de l'appellation « chambres de commerce et d'industrie françaises à l'international » et a pour mission de rassembler, représenter, coordonner et développer le réseau des CCI françaises à l'étranger. Il s'agit aujourd'hui de renforcer son action et ses moyens, pour en faire le véritable bras armé de notre pays à l'international. Dans un contexte économique tendu, la France se doit de conserver un réseau fort à l'étranger pour accompagner nos entreprises, pour favoriser la coopération et le transfert de savoir-faire entre elles, pour poursuivre un travail de structuration et de consolidation des communautés d'affaires à l'étranger et pour développer la formation de ses collaborateurs.

et visant à renforcer la convergence des méthodes du réseau, de recruter des volontaires internationaux en administration pour renforcer les coordinations régionales, de promouvoir la digitalisation du réseau CCI France International à l'étranger et de favoriser la mise en relation des communautés d'affaires.

mise à disposition de locaux ainsi que d'un soutien logistique et administratif, sans parler des missions de formation et d'aide à l'emploi menées auprès des Français de l'étranger et des collaborateurs locaux. Dans un contexte de plus en plus concurrentiel, certains de nos partenaires sont également nos adversaires économiques les plus sérieux, cet amendement vise à renforcer notre réseau afin de lui donner les moyens de se développer. Quel est l'avis de la commission

ne justifie que les crédits de la diplomatie soient mis à contribution pour financer ce qui relève de la politique économique et d'exportation de la France. D'où l'avis défavorable

Quel est l'avis de la commission ? La Caisse des Français de l'étranger est une caisse de sécurité sociale, c'est-à-dire un organisme privé assurant une mission de service public.

Cet amendement vise à doubler les crédits alloués aux organismes locaux d'entraide et de solidarité (Oles). En 2023, 91 associations locales bénéficieront d'une dotation de 1,4 million d'euros, identique à celle de 2022. Nous le savons d'ores et

D'autre part, on peut prévoir que l'extinction du dispositif de secours occasionnel de solidarité, versé par les conseils consulaires pour la protection et l'action sociale pendant la pandémie, entraînera le report des demandeurs d'aide sociale vers les Oles. En outre, il faut anticiper l'inflation et la baisse du cours de l'euro, sur lequel reposent les aides sociales.

Les alliances françaises sont, vous le savez, des associations de droit local privé, autofinancées à 90 % par des cours de français. Elles bénéficient également de subventions publiques pour l'organisation d'événements culturels.

ces organismes ont été fortement affectés par les crises sanitaire et économique. Les confinements ont eu pour conséquence une baisse de leur activité d'enseignement, qui a pesé sur les ressources propres. À cela s'ajoutent des factures énergétiques en hausse, qui risquent d'aggraver des trésoreries déjà fortement fragilisées. Le soutien de l'Institut français, à Paris, ne pourra que renforcer les activités culturelles et l'image des instituts locaux, et attirer de nouveau des publics dont ils ont grand besoin. De plus, depuis la sortie de la pandémie, l'augmentation de la demande dans le secteur culturel et artistique est exponentielle. Les artistes français ont été empêchés de travailler pendant de longs mois. Or, pour beaucoup, aller à l'étranger fait partie de leur mission. Cette subvention exceptionnelle permettrait à la fois d'accroître la visibilité des artistes français à de soutenir l'activité culturelle locale, en mettant en lumière le travail des artistes locaux. La scène française participe, dans le monde entier, à la promotion de nos valeurs, telles que la liberté d'expression et de circulation, dont nous avons grandement besoin aujourd'hui.

La France bénéficie d'un vivier important de volontaires internationaux

très défavorables. Il devient très difficile pour ces VIA de se loger, de se nourrir, de se chauffer, de se déplacer. Certains sont forcés de déménager dans des quartiers lointains, où la sécurité n'est pas optimale,

l'avis de la commission

rectifié. Les conseillers des Français de l'étranger et les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger sont élus au suffrage universel. Ils ne touchent pas d'indemnité, ils sont bénévoles. Seulement, voilà : dans l'exercice de leur mandat, ils supportent évidemment des frais de déplacements, ne serait-ce que pour participer à un conseil d'école dans un lycée français à l'étranger. Une partie modique de ces frais de mandat est couverte.

D'une part, cette situation ne saurait concerner que les conseillers membres de l'Assemblée des Français de l'étranger, puisque les conseillers consulaires disposent, le cas échéant, d'une dotation complémentaire qui permet de rembourser la différence entre les frais de déplacement engagés et un taux forfaitaire fixé par décret. D'autre part, cette situation, si elle existe, doit être relativement marginale. En tout état de cause, elle ne saurait justifier à elle seule d'augmenter de 535 000 euros les crédits dédiés aux indemnités, ce qui correspond à une augmentation de 25 % des crédits demandés. Par ailleurs, les modalités d'indemnisation des conseillers des Français de l'étranger relèvent formellement du domaine réglementaire. Aussi, l'amendement, s'il était adopté,

Renaud-Garabedian. Les Françaises vivant à l'étranger qui sont victimes de violences conjugales ne bénéficient d'aucune aide financière et sont orientées par les consulats vers des structures d'accueil, qui sont liées à des associations.

à l'étranger. Les Françaises qui vivent à l'étranger et qui sont victimes de violences conjugales se retrouvent dans des situations de précarité encore plus importantes que celles qui vivent en France. Quand elles sont mariées à un ressortissant du pays, qui maîtrise le droit, qui est capable de les forcer à rester sur place, qui peut obtenir la garde des enfants si elles n'ont pas accès à un avocat, quand elles ne parlent pas la langue du pays,

nous interrogeons sur les marges de manoeuvre concrètes dont disposent aujourd'hui les postes consulaires pour financer de telles opérations. Les membres de la commission des finances ne sont pas omniscients. Sur cette question, nous sollicitons l'avis du Gouvernement.

notamment à l'allocation à durée indéterminée, qui peut être octroyée à nos ressortissants en difficulté à la suite d'une séparation résultant d'un conflit familial lié ou non à des violences intrafamiliales. Un secours mensuel peut également être accordé aux enfants.

en France et la réinsertion des personnes victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Enfin, pour ce qui concerne la difficulté pour les victimes de financer leur retour en France, le soutien de mon ministère se traduit par la prise en charge financière des titres de transport et des formalités administratives de retour pour la victime, le cas échéant accompagnée de ses enfants, lorsque toutes les autres solutions recherchées ont été infructueuses.

Mme Mélanie Vogel. Cet amendement vise à créer un programme pour accompagner les Français établis hors de France face à la dématérialisation des services consulaires. Ne vous méprenez pas, je ne suis

pour mettre en oeuvre des opérations visant à renforcer l'inclusion numérique des Français établis hors de France. Bien sûr, il peut toujours amplifier ses dispositifs et ses interventions- nous l'invitons d'ailleurs à le faire -, mais, pour ces deux raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. Quel est l'avis du Gouvernement

tous les publics. C'est d'ailleurs ce que nous faisons : d'abord, nous mettons en place de France Consulaire, un service de réponse téléphonique qui se déploie progressivement dans un nombre croissant de pays ; ensuite, un service d'accueil téléphonique et des bornes informatiques sont en place dans de

pratiquer l'IVG pour des raisons religieuses, morales ou autres- je pense en particulier à l'Italie -, ce qui laisse des milliers de femmes dans un état de détresse. Il faut savoir que 72 % des personnes ayant avorté étaient sous contraception et qu'une femme ou personne menstruée sur trois a avorté ou avortera dans sa vie, que ce soit en France ou à l'étranger. Les Françaises qui vivent à l'étranger doivent pouvoir être rapatriées en France en cas d'urgence afin de pouvoir bénéficier de leur droit fondamental à disposer de leur corps. Imaginez qu'on laisse une Française au Brésil à douze semaines de grossesse sans aucune aide et dans l'impossibilité de payer un billet d'avion à un prix exorbitant pour respecter le délai de quatorze semaines. Cela n'est pas acceptable. C'est pourquoi je vous propose de

qui veulent réaliser une IVG, quand ce n'est pas possible dans leur pays de résidence. Je pense que la question doit être prise très au sérieux, en particulier dans

? Les moyens dont disposent les postes diplomatiques pour accompagner les personnes nécessitant un rapatriement d'urgence suffisent-ils ou devraient-ils être abondés sans que soit pour autant créé un programme spécifique

ou de verser une avance remboursable. Pour mémoire, sur la page 32 du passeport français figure ceci : « Les postes diplomatiques et consulaires français ne prennent pas en charge les frais de séjour et de rapatriement. » Je comprends ce qui motive cet amendement, mais il serait particulièrement inéquitable de réserver de nouvelles dispositions aux personnes qui recherchent un rapatriement pour interruption volontaire de grossesse

est possible, bien qu'exceptionnelle, et est décidée après instruction du dossier sur une base individuelle au regard de la situation médicale du patient.

des Français de l'étranger. Enfin, il s'agit d'offrir une cellule d'expertise et d'assistance pour les conseillers des Français de l'étranger. permettra aux élus représentant les Français établis hors de France d'effectuer leur mission de représentation dans de bien meilleures conditions qu'à l'heure actuelle. Quel

Si l'on est gay, lesbienne, bisexuel, transgenre ou intersexe, ce qui est le cas d'un certain nombre de nos compatriotes à l'étranger, on risque des amendes, la prison, des thérapies forcées, de la violence, voire, dans de nombreux pays, la peine de mort.

En Russie, en Pologne, en Hongrie, dans certains États des États-Unis et ailleurs, il est parfois simplement interdit d'évoquer son existence. Cela conduit de nombreux Français vivant hors de France à cacher le fait qu'ils font partie de la communauté LGBTQIA+ afin de ne pas vivre ces discriminations et ces violences. La France se doit de protéger tous ses citoyens et de prendre en compte leurs besoins spécifiques.

la création de la plateforme de réponse aux appels et courriels France Consulaire. Durant la phase d'expérimentation, l'outil semble avoir donné satisfaction, mais il reste perfectible, car le retour d'expérience fait état de certaines réponses inexactes données par les téléconseillers du prestataire,

France Consulaire » pour relater précisément la durée moyenne de réponse aux appels et aux courriels, le taux de transmission des questions au deuxième pôle d'encadrement, ainsi que le taux de satisfaction au regard de l'exactitude des renseignements prodigués. Quel est l'avis de la commission

Conway-Mouret. La réserve parlementaire, qui permettait de venir en aide à des associations à hauteur de 3 millions d'euros, a été remplacée en catimini par le dispositif de soutien au tissu associatif des Français de l'étranger (Stafe). Ce système a vite démontré ses limites, puisque ses crédits, réduits à 2 millions d'euros, n'ont jamais été pleinement utilisés

du nombre de demandes de subvention : il est passé de 368 en 2019 à 242 en 2022. Un groupe de travail sur les critères d'éligibilité au Stafe a été créé avec les conseillers du Français de l'étranger, il s'est réuni une première fois au début du mois de septembre 2022. a pour objet de compléter ce travail, en demandant au Gouvernement de présenter au Parlement un rapport élaboré sur la base des remontées de l'ensemble des conseillers des Français de l'étranger et des associations les représentant. permettrait de clarifier les critères d'éligibilité à ces subventions et de mettre en place un système dans lequel le pouvoir décisionnel revient à ceux qui connaissent le mieux les associations, c'est-à-dire les conseils consulaires.

l'AEFE. Il a suscité une certaine émotion ces dernières semaines et nous proposons de le supprimer pour deux raisons. D'une part, pour une raison de fond nous estimons que le dispositif proposé aurait des effets extrêmement importants sur la gestion de l'enseignement français à l'étranger et sur l'équilibre entre les établissements en gestion directe et l'Agence elle-même.

plus juridique. Ce dispositif se borne à réviser les modalités de la gouvernance de l'AEFE et de ses relations financières avec les établissements.

à emprunter pour financer ses investissements immobiliers. À cela s'est ajoutée en 2017 la suppression de la garantie de l'État ; c'est donc la double peine ! Pour accueillir davantage d'élèves, comme le souhaite le Président de la République, les établissements auront besoin d'ouvrir des classes et donc d'agrandir les bâtiments.

d'ordre général. Les crédits demandés- environ 8 milliards d'euros en autorisations d'engagement et 5,9 milliards d'euros en crédits de paiement -ne représentent qu'une partie de l'aide publique au développement. En 2022, la France se situe au cinquième rang des pays donateurs après les États-Unis, l'Allemagne, le Japon et le Royaume-Uni. Le montant global de l'aide, qui s'élève à 13,1 milliards d'euros, représente

Il nous faudra sans doute revoir cet objectif, devenu trop ambitieux au regard des contraintes qui pèsent désormais sur nos finances publiques. En effet, pour atteindre un tel niveau, nous devrions accroître l'aide publique au développement de 10 milliards d'euros en deux ans, ce qui semble trop élevé.

En ce qui concerne les pays bénéficiaires, l'aide publique au développement de la France est principalement tournée vers l'Afrique. Je profite de cette occasion pour indiquer que, désormais, la France n'engage la France n'engage plus de crédits comptabilisés comme de l'aide publique au développement en Chine, comme c'était encore le cas naguère. De plus, si la Turquie perçoit 41,4 millions d'euros, il s'agit de crédits versés pour financer le mécanisme d'accueil des réfugiés syriens. Vous le savez, le principal opérateur de l'aide publique au développement en France est l'Agence française de développement (AFD), dont le portefeuille d'activités correspond à un montant d'environ 12 milliards d'euros. Cet opérateur ne perçoit pas de subventions de fonctionnement de la part de l'État, mais il perçoit des crédits qui compensent à la fois la part concessionnelle des prêts accordés et les subventions versées sans contrepartie. L'AFD et ses tutelles négocient en ce moment le prochain contrat d'objectifs et de moyens (COM), dont l'un des buts principaux sera de resserrer le nombre des indicateurs de suivi, afin de rendre le pilotage plus stratégique ; cette idée nous semble intéressante. Par ailleurs, notre rapport présente pour la première fois quelques développements sur l'aide engagée par les collectivités territoriales. Si elle reste encore modeste, avec un montant d'environ 145 millions d'euros, cette aide est en progression depuis 2018. Mon collègue Jean-Claude Requier, qui va me succéder à cette tribune, dira quelques mots pour présenter plus précisément les crédits des programmes qui composent cette mission et le compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers Toutefois, je souhaite vous rappeler qu'au nom de la commission des finances nous porterons un amendement visant à réduire de 200 millions d'euros crédits de la mission « Aide publique au développement

économiques (OCDE), ne peut pas être liée à l'obtention de faveurs de la part des États que nous aidons. Le contexte budgétaire qui est le nôtre nous oblige à prioriser nos efforts afin de privilégier nos concitoyens et nos intérêts en tant que puissance. Pour cette raison, si nous devons préserver les moyens de la sécurité, de la défense, de la diplomatie, de la santé et de l'éducation, nous devons en tirer les conséquences sur l'ampleur de la politique de solidarité que nous menons à l'égard du reste du monde.

En 2023, ce budget augmente très fortement. En effet, les autorisations d'engagement connaissent une hausse de 1,4 milliard d'euros et les crédits de paiement de plus de 819 millions d'euros. Le programme 209, « Solidarité à l'égard des pays en développement », qui relève du ministère des affaires étrangères, concentre les hausses les plus importantes. Ainsi, le montant des crédits demandés augmente de 837 millions d'euros en autorisations d'engagement et de 383,1 millions d'euros en crédits de paiement, afin notamment de renforcer les capacités de gestion de crise et de soutenir les politiques de santé au niveau mondial, comme cela était déjà le cas en 2022. En matière de santé, les crédits augmentent de 336,4 millions d'euros en autorisation d'engagement, en raison de la mobilisation de 256,7 millions d'euros pour la reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, et du financement consacré à l'alliance Gavi, à hauteur de 94,7 millions d'euros. Par ailleurs, la création d'un mécanisme de réserve pour les crises majeures explique une hausse de 270 millions d'euros des crédits demandés sur ce programme. Cette enveloppe viendra compléter les 460 millions d'euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement déjà consacrés aux opérations de gestion et de sortie de crise. La création de ce mécanisme de réserve paraît bienvenue, puisqu'elle permettra de donner aux responsables de programmes des marges de manoeuvre pour financer des dispositifs d'urgence sans mettre en cause le financement d'opérations déjà engagées. Toutefois, nous nous interrogeons sur les garanties qui seront apportées par le Gouvernement pour que ces crédits ne constituent pas une réserve de budgétisation par temps calme et qu'ils donnent bien lieu à des annulations ou à des reports en fin de gestion. En outre, nous estimons que le montant demandé est relativement élevé compte tenu des autres crédits disponibles pour faire face à l'urgence. Pour cette raison, et afin de financer les mesures d'économies demandées à la mission, l'amendement de la commission des finances, que nous présenterons tout à l'heure, vise à diminuer de 100 millions d'euros les crédits de cette enveloppe. Sur le programme 110, qui, lui, relève du ministère de l'économie et des finances, le montant des crédits demandés pour 2023 connaît une forte augmentation, de 632 millions d'euros en autorisations d'engagement et de 475 millions d'euros en crédits de paiement. Cette hausse s'explique surtout par la persistance d'un important besoin de crédits pour participer aux cycles de refinancement des fonds internationaux. Par ailleurs, les effets de la hausse des taux d'intérêt sur le coût des opérations de sur le coût des opérations de bonification de prêts jouent aussi un rôle. En effet, afin de permettre à l'AFD de prêter à des taux concessionnels aux bénéficiaires de l'aide au développement, l'État prend en charge, par le versement de crédits de bonification, la différence entre le coût de financement de l'AFD et le taux auquel elle prête à ces pays. Or, dans le contexte de remontée des taux d'intérêt mondiaux, les coûts de financement de l'AFD ont augmenté, alors même que, pour être considérés comme concessionnels, les taux proposés doivent rester inférieurs à un seuil fixé par l'OCDE. Ainsi, afin de maintenir le niveau d'aide publique au développement permis par les prêts de l'AFD, le ministre de l'économie et des finances a pris la décision d'accroître le montant des crédits affectés à la bonification des prêts de 390 millions d'euros en 2023. des crédits importants sont demandés au titre du programme 110, afin de participer à la reconstitution des ressources de divers fonds internationaux, tels que le Fonds vert pour le climat. Enfin, le programme 365 est consacré à la recapitalisation de l'AFD. Comme l'année dernière, les 190 millions d'euros demandés correspondent à une opération de conversion de ressources financières de l'AFD en crédits budgétaires. Cette opération est totalement neutre pour les finances publiques en comptabilité nationale. Il ne s'agit ni d'accroître les engagements de l'État envers l'AFD ni de lui permettre d'augmenter son volume d'activité, figé à 12 milliards d'euros. Comme l'a indiqué notre collègue Michel Canévet, sous réserve de l'adoption de l'amendement que nous vous présenterons, la commission des finances, par la voix de ses rapporteurs spéciaux, vous invite à adopter les crédits de la mission « Aide publique au développement » et ceux du compte de concours financiers

D'un côté, cette hausse reflète la volonté, manifestée à l'unanimité lors du vote de la loi du 4 août 2021, de faire de la solidarité internationale une composante à part entière de notre action extérieure, au même titre que notre diplomatie et notre défense. La finalité en est simple : lutter de manière préventive contre les causes profondes des désordres mondiaux que sont les crises, les conflits ou encore les déplacements de populations. La progression des crédits en dons de l'Agence française de développement permettra ainsi de renforcer cette indispensable politique de solidarité internationale. Concrètement, ce sont des crédits supplémentaires pour l'éducation, pour la santé, ou encore pour l'agriculture, avec une concentration sur les pays d'Afrique subsaharienne. D'un autre côté, la progression des crédits est aussi à la mesure d'une situation mondiale qui se dégrade fortement, avec de multiples crises politiques, sociales et alimentaires, de l'Afrique subsaharienne à l'Afghanistan, en passant par le Moyen-Orient. D'où la forte augmentation de l'enveloppe budgétaire « Gestion et sortie de crise », qui passe de 297 millions en 2022 à 730 millions d'euros en 2023. Il s'agit d'un effort de rattrapage salutaire, car, malgré cette évolution considérable, la France ne figure qu'au septième rang des vingt-sept bailleurs européens. Il faut souligner que nos instruments d'aide humanitaire et d'aide au développement sont également mis en oeuvre en Europe dans la crise actuelle. dans la crise actuelle. Outre notre aide humanitaire, l'Ukraine a ainsi bénéficié d'un prêt de 300 millions d'euros de l'AFD dès avril 2022. Il faut se féliciter de cette réactivité, qui montre que l'Agence peut être un instrument politique capable de mettre en oeuvre rapidement les priorités du Gouvernement. L'AFD a d'ailleurs également apporté une aide significative à la Moldavie. Les crédits en hausse nous permettront donc de poursuivre ce soutien aux États européens agressés par la Russie. L'augmentation de ces différents budgets peut paraître excessive à un moment où il nous est demandé de faire des économies, mais la politique d'aide au développement est un élément majeur de notre action extérieure et de l'influence française. Son rôle premier est, certes, de venir en aide et au soutien de peuples défavorisés, mais elle a aussi pour objectif objectif d'offrir des perspectives locales là où l'aspiration des populations est de rejoindre nos économies pourtant fragilisées. Au total, ce budget de l'APD pour 2023 devrait donc permettre à notre pays de montrer son meilleur visage sur la scène internationale. le réduire considérablement serait révélateur d'une vision étriquée là où nous devons, au contraire, nous déployer. Au moment où nos adversaires attaquent notre image par tous les moyens et sur tous les continents, l'APD nous donne un point d'appui pour développer un contre-discours offensif. Cette approbation globale ne doit cependant pas nous empêcher d'être vigilants sur certains sujets, en particulier la mise en oeuvre complète des orientations de la loi du 4 août 2021, qui sera évoquée plus précisément par mon collègue rapporteur pour avis

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues,

je veux insister sur la gouvernance. Nous lançons là un véritable SOS pour le comité interministériel de la coopération internationale et du développement (Cicid), tant de fois annoncé, mais jamais réuni depuis février 2018. Cette situation est inacceptable et elle empêche toute discussion parlementaire sur le contrat d'objectifs et de moyens de l'AFD pour la période 2023-2025. Rappelons que le dernier COM a été validé six mois avant la fin du précédent ailleurs, je m'interroge sur des dispositions qui sont au coeur de la volonté du législateur et dont l'application est encore parfois « brumeuse ». Je pense par exemple aux droits et à la protection de l'enfance, disposition législative, qui, je le rappelle, n'est pas une option. Je pense aussi aux objectifs fixés en matière de rapport dons-prêts, de part d'aide bilatérale et de concentration de l'aide programmable sur les pays prioritaires le compte n'y est toujours pas. Nous regrettons également que, cette année encore, moins d'un tiers de la taxe sur les transactions financières soit consacré au développement, qui est pourtant la raison d'être de cette taxe.

le programme 110, « Aide économique et financière au développement », placé sous la responsabilité du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ; le programme 209, « Solidarité à l'égard des pays en développement », qui, lui, est piloté par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Conformément à la trajectoire financière tracée, les crédits de paiement affectés à ces deux programmes sont en augmentation de plus de 17 % par rapport à la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 et atteignent 5,9 milliards d'euros. Cette augmentation, qui intervient dans une période post-crise sanitaire, durant laquelle la maîtrise des dépenses de l'État est redevenue une priorité, témoigne de la volonté de la France de rester un soutien fort et fiable des pays en voie de développement. Ce choix est rendu nécessaire par le contexte international, mais c'est aussi un choix politiquement courageux au regard du contexte politique national que l'on connaît. Oui, la France a ses propres enjeux, ses propres urgences et, sans doute,

non pas simplement d'approuver l'augmentation des crédits de l'APD, mais de la revendiquer. La hausse de 46 % de l'aide économique et financière au développement va permettre à la France de continuer à accorder des taux d'emprunt très bas aux pays en développement. Certains reprochent au Gouvernement ce choix de préférer les prêts plutôt que les dons ou les subventions, mais il importe de responsabiliser les États, car il n'y a pas d'« argent magique », pour reprendre une formule du Président de la République. autant, l'engagement de la France dans l'aide internationale doit rester financièrement soutenable. Le périmètre « OCDE » de l'APD s'élève en 2022 à 14,8 milliards d'euros, soit à environ 0,55 % du revenu national brut. Soyons réalistes

Cela n'enlève rien à la volonté de contribution de la France, comme en témoigne la hausse spectaculaire des crédits de « gestion et sortie de crise », qui passent à 730 millions d'euros, soit une augmentation de 146 %. Voilà un chiffre éloquent ! Il faut aussi souligner l'augmentation des fonds consacrés à l'aide humanitaire, qui atteignent 642 millions d'euros, contre 500 millions d'euros l'an passé. Soyons donc fiers de ce budget, qui est, certes, davantage tourné vers l'aide humanitaire que vers le développement, mais qui a le mérite de s'adapter véritablement aux besoins de l'instant. Notre aide humanitaire programmée va en effet atteindre 635 millions d'euros : 200 millions d'euros mis en oeuvre le fonds d'urgence et de stabilisation, notamment pour l'Irak- je m'en réjouis en tant que présidente du groupe d'amitié France-Irak -, mais aussi pour la Syrie, la Libye, le Yémen, l'Afghanistan ou encore la zone subsaharienne pour l'aide alimentaire programmée ; 200 millions d'euros affectés aux contributions humanitaires volontaires aux Nations unies ; 75 millions d'euros pour le (Farm), qui doit répondre spécifiquement aux problèmes alimentaires mondiaux provoqués par le conflit ukrainien. Autant d'efforts budgétaires qui permettent à la France d'occuper la septième place parmi les vingt-sept pays de l'Union européenne en matière d'aide humanitaire. Pour que la France maintienne un niveau d'engagement qui lui permette de peser dans les arbitrages et de faire entendre sa voix dans le concert européen et international, le groupe RDPI est favorable à l'adoption des crédits de cette

d'État, mes chers collègues, l'aide publique au développement est un pilier de la politique étrangère de la France et contribue à assurer la paix et la sécurité dans le monde. Cette définition résulte de la loi du 4 août 2021 relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, pour laquelle le Sénat, et plus particulièrement les membres de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées,

bien que notre groupe eût souhaité, sur beaucoup de points, une position plus ambitieuse. Cette loi propose notamment la création d'un mécanisme de restitution des biens mal acquis. Les socialistes ont beaucoup oeuvré dans ce sens et je tiens tout particulièrement à rendre hommage au travail réalisé sur cette question par notre collègue Jean-Pierre Sueur. Bien d'autres engagements ont été pris dans cette loi. Nous attendons désormais que chacun d'entre eux soit suivi d'effet ... Sur la trajectoire financière de l'aide publique au développement, une position de compromis avait été trouvée lors des débats. Nous souhaitons que celle-ci soit

C'est un combat que nous rappellerons chaque fois que le débat le permettra. Si l'Agence française de développement a pour mission de financer des projets de développement par des dons, elle accorde également une grande part de ses financements au travers de prêts bancaires.

de nombreux pays qui bénéficient de prêts se trouvent dans des situations proches du surendettement. Nous regrettons qu'une fois de plus le projet de loi de finances ne rééquilibre pas la part entre ces deux piliers : les prêts et les dons. La solidarité française ne doit pas être monnayée. La situation économique mondiale plaide, plus que jamais, pour l'octroi de dons plus importants. L'aide publique au développement a aussi pour objectif d'éradiquer la pauvreté, de lutter contre les inégalités, de promouvoir les droits humains et de renforcer l'État de droit. À nos yeux, la promotion de l'enregistrement des naissances et la mise en place d'états civils fiables doivent être une priorité de la politique de développement solidaire de la France.

En 2019, un rapport de l'Unicef soulignait qu'un enfant de moins de 5 ans sur quatre n'était pas enregistré à la naissance et que ce ratio s'accentuait en Asie du Sud et en Afrique. Pour ces enfants, qui deviendront des adultes invisibles, sans état civil, il n'y aura aucun accès aux droits les plus élémentaires. Ils seront à la merci de trafics en tout genre, des mariages forcés, de la prostitution. Nous attendons de la France qu'elle ait une position ambitieuse dans la promotion de la constitution d'états civils fiables, qu'elle contribue au fonds du groupe de travail pour l'identité juridique et nous entendons que le Gouvernement consente enfin à nous communiquer le montant de sa contribution.

Ce pays, qui fut un modèle de démocratie en Afrique, vit aujourd'hui une situation très grave. La junte met en scène le rejet de la France, manipule ses opinions publiques et laisse des pans entiers de son pays aux mains des terroristes ou des milices de Wagner.

? Cette situation nous inquiète doublement, d'autant que le gouvernement malien, même s'il est peu crédible, a, en guise de réponse, déclaré « interdire, avec effet immédiat, toutes les activités menées par les associations, les organisations non gouvernementales et assimilées opérant sur le territoire de la République du Mali, sur financement ou avec l'appui matériel ou technique de la France D'une part, nous ne serons jamais favorables à la rupture de tout lien avec des associations engagées sur le terrain, sur des projets qui contribuent le plus souvent à maintenir à flot un embryon de démocratie. D'autre part, de nombreuses collectivités territoriales s'interrogent sur le futur de leur coopération décentralisée. Elles ont besoin d'être éclairées, voire confortées. Mesdames les ministres, je souhaite que ce débat vous donne l'occasion de nous apporter toutes les réponses

madame la ministre, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, cette année, le budget de l'aide publique au développement augmente de 800 millions d'euros. Nous progressons, certes, mais lentement, trop lentement, au point de repousser dès cette année l'objectif de 0,7 %, faute d'avoir pu

contenus trop souvent conçus non pour aider les pays destinataires à s'émanciper durablement de leurs dépendances, mais d'abord pour préserver les intérêts français dans les régions concernées.

ceux qui en ont le plus besoin, tandis que certains pays plus riches et mieux dotés en DTS ne les utilisent pas tous. Une autre injustice continue de nous scandaliser. Alors que le produit de la taxe sur les transactions financières

de l'aide publique au développement, pour servir à rembourser une dette créée par notre pays. L'argent ira donc dans la poche de créanciers qui vivent des intérêts de cette dette,

alors que, pour la première fois depuis 1990, l'extrême pauvreté augmente et que l'indice de développement humain global diminue pour la deuxième année consécutive. Madame la ministre, comment peut-on continuer à justifier

mais aussi en France. Faire ainsi payer les frais des désaccords politiques entre nos deux gouvernements à l'une des populations les plus pauvres du monde, c'est une faute !

Avec ce projet de loi de finances, l'objectif, annoncé par le Président de la République en 2017, de porter à 0,55 % la part de notre revenu national brut consacrée à l'aide publique au développement est atteint. Nous avions entériné cet objectif l'an dernier, au travers de la loi du 4 août 2021 ; nous saluons donc le respect de cet engagement. La cible de 0,7 % du RNB, fixée depuis 1970 par l'ONU, sera quant à elle repoussée de 2025 à 2030 en raison de la crise économique

Ces crédits vont permettre une action approfondie dans les trois zones de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et du Sahel. En tant que président du groupe interparlementaire d'amitié France-Afghanistan et que membre du groupe France-Ukraine, je ne peux que souscrire à la création d'enveloppes dédiées à ces deux pays qui se trouvent dans des situations extrêmement difficiles. Dans le cadre de la guerre en Ukraine, l'Agence française de développement apporte sa pierre à l'aide humanitaire, mais aussi à l'aide au développement, non seulement en Ukraine, mais encore en Moldavie et en Roumanie. Cette adaptabilité du groupe AFD aux changements de contexte international doit être soulignée ; nous ne pouvons que nous en féliciter. Plus largement, ce sont tous les crédits de la mission qui augmentent en 2023, avec 1,4 milliard d'euros supplémentaires en autorisations d'engagement et 819 millions en crédits de paiement. Cette augmentation correspond aux ambitions et orientations fixées l'an dernier dans la loi de programmation de notre aide publique au développement.

où il s'élevait à 60 %. Le report de la cible de 0,7 % du RNB, évoqué au début de mon intervention, pose également question : le Parlement sera-t-il associé à la réactualisation nécessaire de la programmation financière prévue par la loi ? De la même manière, la création, dans ce projet de loi de finances, d'un mécanisme de réserve pour crise majeure, doté de 270 millions d'euros, est bienvenue pour renforcer le dynamisme et la réactivité de l'aide humanitaire française, mais ce mécanisme ne doit pas devenir une réserve de budgétisation. La loi de programmation a également mis en avant le besoin de transparence de notre aide au développement. Nous nous réjouissons donc de la récente mise en ligne, par le ministre de l'économie et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, d'une base de données ouvertes visant à regrouper les informations relatives à l'APD de notre pays. Ce travail sur la transparence a déjà été reconnu par le gain de cinq places enregistré par l'AFD dans le classement de l'ONG, qui analyse la qui analyse la transparence des principales agences de développement dans le monde. En revanche, il faut tout de même souligner que la mise en place de la commission d'évaluation de l'aide alors qu'elle doit devenir un véritable instrument de transparence et d'efficacité de notre politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. ! Alors que la France vit une crise d'influence, notamment en Afrique, continent prioritaire de notre politique de développement, il est nécessaire de renforcer encore davantage cette transparence. Il est aussi indispensable de mettre en avant notre politique de développement et notre apport à la solidarité internationale par des actions de communication à destination des populations bénéficiant des projets, notamment les jeunes générations. L'augmentation de l'aide bilatérale doit aller de pair avec une lutte contre la désinformation à l'encontre de la France. Cette affirmation est particulièrement vraie au Sahel, où la stratégie 3D- défense, diplomatie, développement -a mal fonctionné, notamment en matière de coordination entre la défense et le développement, et où nos efforts politico-militaires ont été refoulés, comme l'illustre aujourd'hui la crise profonde avec les autorités maliennes. Le 16 novembre dernier, tous les projets de développement français ont été suspendus au Mali, pour éviter tout risque de détournement. On peut s'interroger sur la suite des événements : que vont devenir les projets en cours et les financements prévus Le Sénat restera attentif aux orientations données à la politique de développement française, tout particulièrement lors de la prochaine réunion du comité interministériel de la coopération internationale et du développement, qui devrait se tenir au début de l'année prochaine.

Sans renoncer à notre politique d'influence humanitaire à l'étranger et à un nécessaire à la française, nous devrions ajuster ce budget au contexte national de tension financière exceptionnelle. Il m'est impossible de soutenir le projet contesté d'un nouveau siège pour l'Agence française de développement, qui coûterait 1 milliard d'euros au contribuable français. Cette somme, c'est précisément ce qu'Emmanuel Macron a refusé d'investir en 2019 pour financer le nucléaire du futur, sacrifiant ainsi notre indépendance énergétique Je dénonce également les 41 millions d'euros versés à la Turquie dans le cadre du mécanisme d'accueil des réfugiés syriens, alors que le sultan Erdogan ne se prive pas de faire du chantage aux clandestins à nos frontières européennes et de soutenir l'invasion de l'Arménie par l'Azerbaïdjan. Par ailleurs, je vois mal l'intérêt de financer de l'aide humanitaire dans un Afghanistan totalement sous l'emprise des talibans, car nous n'avons aucun contrôle sur la destination de ces fonds. Cependant, nous ne devons pas seulement nous demander combien nous dépensons, mais aussi comment nous dépensons. En effet, le retour sur investissement de cette dépense publique est gravement mis en cause. Pour avoir tiré la sonnette d'alarme chaque année, je peux vous dire que je regrette chaque euro dépensé pour le Mali, qui nous aura offert en retour la haine, la haine, de sa population comme de son gouvernement, à l'égard de la France. Cela doit nous servir de leçon ! L'aide publique au développement doit être conditionnée à nos intérêts, afin de garantir la sécurité de notre territoire en contrôlant les trafics et les flux humains bien en amont. Elle doit être conditionnée à l'acceptation automatique, par les États bénéficiaires, de leurs étrangers expulsés de notre territoire national. N'ayant pas de consignes claires quant à la conduite à tenir, l'AFD ne se soucie pas de soutenir les entreprises et l'industrie françaises lorsqu'elle finance un projet à l'étranger. C'est tout à fait déplorable En outre, le Président de la République vient de déclarer que la France allait débloquer une enveloppe de 1 milliard d'euros pour aider l'Afrique du Sud à sortir du charbon, alors que les choix de ce même Président ont entraîné la réouverture de centrales à charbon sur notre sol. Regardons la poutre qui est dans notre oeil plutôt que le charbon dans celui du voisin ! Il y a tant à faire dans notre pays en matière de développement ... Il faut que chaque euro dépensé à l'étranger serve au développement du pays en savoir-faire et en infrastructure, afin que les populations se fixent, deviennent autonomes et prospèrent.

mes chers collègues, cette mission s'inscrit au coeur des valeurs que la France défend, celles de solidarité et de respect des droits humains, des valeurs que tous En tant que pays développé, pour ne pas dire riche, nous avons le devoir de préserver une aide au développement ambitieuse, en faveur du droit à une vie digne pour tous. rapporteurs spéciaux ont exposé les chiffres qui confirment la hausse du soutien de la France : les crédits de la mission « Aide publique au développement » augmenteront de 16,04 % en 2023. Avec un montant total d'aide de 14,8 milliards d'euros selon les critères de l'OCDE, on peut se réjouir que notre pays ait rempli, en 2022, son objectif d'une aide portée à 0,55 % du revenu national brut, conformément à la loi de programmation du 4 août 2021. 2021. Toutefois, comme pour les autres missions budgétaires, l'inflation, hélas ! imprime sa marque. En effet, en raison de la situation économique actuelle, l'objectif de 0,7 % du RNB est reporté de 2025 à 2030. C'est bien entendu regrettable, mais on peut espérer qu'il sera possible de réinscrire, au plus vite, nos moyens dans une trajectoire plus dynamique. En attendant, il me semble essentiel que les crédits proposés se concentrent sur les zones prioritaires définies par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement en 2018 et réaffirmées depuis lors. À cet égard, madame la ministre, notre politique de développement solidaire est-elle bien concentrée sur les 19 pays prioritaires identifiés, quasiment tous situés en Afrique ?

C'est le choix de la France, que mon groupe partage. Cela dit, ne cachons pas que certains de ces choix sont parfois amers. Je pense à ce qui se passe au Mali, pays dans lequel l'image de la France est injustement abîmée. Il convient toutefois de ne pas renoncer. Ne mettons pas en avant nos liens passés avec le continent africain, ce qui a parfois tendance à irriter. Voyons plutôt l'Afrique pour ce qu'elle est aujourd'hui : le coeur de tous les défis, démographiques, économiques et climatiques. C'est un continent où les vulnérabilités socio-économiques sont structurelles dans la plupart des États. Néanmoins, beaucoup de pays africains ont une formidable capacité de résilience, similaire à celle que l'on observe actuellement au Bangladesh. C'est dans un esprit de partenariat que nous devons accompagner ces pays dans leur développement, sur le fondement d'une coopération plus moderne, qu'il faut sans doute mieux expliquer aux populations, à l'aide de nos outils d'influence. L'urgence, aujourd'hui, c'est de ne pas laisser ces populations s'enfoncer dans la crise alimentaire. L'agression russe en Ukraine a créé une situation dramatique, en particulier au Sahel et dans la Corne de l'Afrique. Je salue donc la hausse des crédits destinés à l'aide alimentaire au sein de cette mission. Enfin, mes chers collègues, je rappelle que faire preuve de solidarité pour le développement, ce n'est pas faire oeuvre de charité. C'est une responsabilité que nous avons en tant que pays du Nord, eu égard à notre modèle de développement qui- il faut bien le dire -a mis la planète en danger. Aussi, je me réjouis de l'avancée de la COP27 la COP27 sur le fonds « pertes et dommages » destiné aux pays du Sud touchés par les dégâts dus au dérèglement climatique. Le RDSE compte sur vous, madame la ministre,

Pandémie de covid-19 ; changement climatique accéléré ; insécurité alimentaire grandissante ; terrorisme ; guerres et regain des tensions internationales ; choc énergétique ; surendettement ; inflation la liste des crises qui secouent le monde ces dernières années semble ne pas devoir s'arrêter de croître. Inévitablement, leurs conséquences humaines s'alourdissent et rendent plus que jamais nécessaire l'aide internationale en faveur des pays les plus fragiles. La France, qui se classe au cinquième rang mondial des bailleurs de fonds, a d'ailleurs consenti depuis dix ans des efforts considérables pour se hisser à la hauteur cet enjeu. Souvenons-nous qu'en 2014 le volume global de ses engagements au titre de l'aide publique au développement était de 8 milliards d'euros, soit 0,37 % de son revenu national brut. En 2022, il est passé, selon nos rapporteurs spéciaux, à 13 milliards d'euros, soit 0,51 % du RNB. L'année prochaine, cette montée en puissance sera une nouvelle fois intensifiée pour dépasser les 15 milliards d'euros et s'établir à 0,55 % du RNB. Les crédits de la mission budgétaire « Aide publique au développement » ne constituent qu'une partie, certes substantielle, de ce vaste ensemble. Pour 2023, le Gouvernement propose de les augmenter de manière très appréciable : la hausse est de quelque 16 % en crédits de paiement.

En effet, les pays les plus fragiles sont largement, voire parfois totalement dépourvus des moyens nécessaires pour amortir les effets des crises. Leurs populations, qui sont déjà les plus vulnérables, sont donc, de fait, les plus menacées. Les soutenir face aux soubresauts qui agitent le monde, comme nous le faisons par exemple en Ukraine, est donc une exigence morale à laquelle nous ne pouvons nous soustraire. Mais permettez-moi, mes chers collègues, de souligner qu'il s'agit aussi de notre intérêt. Dans une économie globalisée, la prospérité des uns ne peut aller durablement de pair avec la paupérisation des autres. En stimulant la vitalité économique des pays en développement

sous-estimons pas le fait que l'aide au développement est également une contribution apportée à la sécurité internationale. C'est particulièrement vrai en Afrique subsaharienne, qui est à la fois la zone d'action prioritaire de l'AFD et le théâtre principal des opérations extérieures que nous avons engagées au cours Y aider les populations à satisfaire leurs besoins fondamentaux- se nourrir, se soigner, s'éduquer -et contribuer à ce qu'elles bénéficient de perspectives économiques, c'est en partie assécher le terreau sur lequel se développent les mouvements djihadistes, contre lesquels nos soldats continuent de lutter. C'est aussi, ne l'oublions pas, contribuer à dessiner un avenir qui ne passe pas automatiquement par les routes migratoires. Au moment où l'opération Barkhane s'achève officiellement, de nombreux enseignements doivent toutefois être tirés de l'action de notre pays dans la région.

Face à ce recul, qui ne cesse de s'accélérer, la redéfinition d'une politique africaine globale est désormais urgente. Elle devra nécessairement inclure une nouvelle réflexion sur les résultats de la politique d'aide au développement que nous y menons. C'est d'autant plus essentiel que le volume, les modalités et les objectifs de l'aide économique revêtent une dimension stratégique qui ne fait que s'affirmer. Cette aide est devenue, en particulier sur le continent africain, un enjeu à part entière dans la lutte d'influence à laquelle se livrent les grandes puissances, dont certaines ne ménagent pas leurs efforts pour nous concurrencer, voire nous évincer. Une aide au développement revisitée doit donc nous permettre de retrouver, dans cette partie du monde, les leviers d'action qui nous échappent peu à peu. Voilà, brossées à grands traits, les raisons qui amènent notre groupe à soutenir, malgré l'extrême difficulté du contexte économique, un nouveau renforcement des crédits de la mission « Aide publique au développement ». aide, c'est une réponse aux risques créés par des crises qui se multiplient et se combinent. Cette aide, c'est aussi un instrument du rayonnement et de l'influence de la France. Cette aide, c'est enfin l'expression des orientations définies dans la loi de programmation du 4 août 2021,

Concernant l'annuité qui nous intéresse aujourd'hui, celle de 2023, la cible initialement fixée à 0,61 % du RNB a en conséquence été ramenée à un niveau plus soutenable de 0,55 %. La dégradation importante de nos comptes publics, l'impact de l'inflation et le risque de récession, de plus en plus prégnant, ne laissaient, à la vérité, pas d'alternative. Il n'en reste pas moins que le Gouvernement propose, en crédits de paiement, de mobiliser 818 millions d'euros supplémentaires au bénéfice de cette mission, qui disposerait ainsi de 5,9 milliards d'euros au total Cette augmentation s'inscrit dans un cadre général, que le Gouvernement a exposé dans son projet de loi de programmation des finances publiques. Or la majorité sénatoriale a contesté, il y a un mois, l'économie générale de ce texte, estimant qu'il ne permettrait pas de réduire le déficit public dans des délais satisfaisants. Le budget général

C'est pourquoi, dans le cadre d'une approche globale et cohérente, notre groupe proposera, par voie d'amendement, de fixer leur progression à 618 millions d'euros l'année prochaine. Il s'agit, nous semble-t-il, d'une voie équilibrée, qui permet de satisfaire à deux exigences en apparence peu conciliables d'un côté, réaffirmer notre engagement à faire plus pour la solidarité internationale, de l'autre, agir résolument pour restaurer la responsabilité et la crédibilité budgétaires de notre pays. La parole

Elle y consacre des sommes importantes, pour améliorer le sort des pays les moins avancés. Cette aide fait une énorme différence pour ceux qui la reçoivent. C'est évidemment le cas de l'aide d'urgence : délivrée dans un contexte de crise humanitaire, elle permet de sauver des vies. Dans des contextes moins tendus, l'aide permet à des populations d'améliorer leurs conditions de vie en construisant des infrastructures essentielles. Enfin, l'aide de la France permet à de nombreux pays de développer leur économie en encourageant la création d'entreprises. Cette aide est bien plus que de la philanthropie, dans la mesure où elle contribue à la sécurité des populations. Les zones les plus défavorisées sont en effet les plus sujettes au développement de conflits armés. Ceux qui n'ont rien n'ont rien à perdre ! Si cette action est utile et si elle est tout à l'honneur de notre pays, elle a un coût. En 2022, la France lui a consacré 13 milliards d'euros, soit 0,51 % de son revenu national brut. Il s'agit d'un effort important, particulièrement dans un contexte économiquement difficile. cinquième contributeur mondial à l'aide au développement, elle n'est plus la cinquième puissance économique. Devancés par l'Inde, nous sommes à présent septièmes. Alors que nous visons toujours l'objectif de consacrer 0,7 % de notre RNB à l'aide au développement, la question des moyens se pose. Michel Canévet, il sera très difficile d'atteindre cet objectif. La plupart des économistes s'accordent à dire que la croissance mondiale sera faible dans les années à venir. La France sera, elle aussi, confrontée à de sérieuses difficultés économiques : très endettée, elle est particulièrement affectée par la remontée des taux d'intérêt. La question de la soutenabilité de cette aide se pose donc, mais on peut aussi s'interroger sur les objectifs de l'aide apportée par la France. Nous avons été plusieurs à souligner que cette aide doit être destinée aux pays qui en ont le plus besoin. Elle doit aussi être orientée vers des projets qui servent nos intérêts. des dernières années, la France a fait l'objet de campagnes hybrides visant à nuire à son image. Force est de constater que ces campagnes ont eu un certain effet ... Il nous paraît essentiel que l'aide publique au développement financée par le contribuable français fasse l'objet d'un contrôle strict et n'aille pas renforcer la gouvernance de pays qui font montre d'hostilité à l'égard de la France. Au côté de l'État, nos collectivités territoriales contribuent de plus en plus à l'aide publique apportée par notre pays. Elles le font, notamment, au travers de projets centrés sur leurs compétences, comme la gestion de l'eau. Les collectivités consacrent également

La France, dans toutes ses composantes, contribue donc beaucoup à l'aide au développement. Elle doit continuer de le faire, selon ses moyens et au bénéfice de projets qui servent ses intérêts. C'est pourquoi le groupe Les Indépendants - République et Territoires votera en faveur de l'adoption des crédits de cette mission. La parole est

Même si la marche est haute, la France doit tout faire pour tenir cet objectif qui, rappelons-le, est une promesse non tenue depuis plus d'un demi-siècle ; il convient, à tout le moins, de s'en approcher au plus près. près. Au vu du contexte géopolitique et économique qui succède à la pandémie, ne tenons pas rigueur au Gouvernement de ne pas avoir respecté cette trajectoire. En effet, l'augmentation brute de 1,4 milliard d'euros en autorisations d'engagement et de 819 millions d'euros en crédits de paiement constitue déjà un signal positif.

Le programme 209 relatif à la solidarité avec les pays en développement augmente de 433 millions d'euros, dont 270 millions d'euros consacrés à la création d'un fonds d'urgence pour faire face aux crises : cela semble particulièrement opportun dans le climat actuel.

Je m'oppose d'ailleurs avec force à leur amendement visant à réduire de 200 millions d'euros les crédits du programme 209. Nous sommes déjà en retard par rapport à la trajectoire budgétaire que la Haute Assemblée a adoptée à la quasi-unanimité : il serait totalement incohérent de réduire l'enveloppe aujourd'hui. Je salue, en revanche, la priorité accordée, dans les actions de la mission, aux besoins prioritaires que sont l'éducation et la santé, avec des augmentations de crédits de 122 millions et 336,4 millions d'euros destinées à respecter les engagements de la France pour le partenariat mondial pour pour l'éducation et à reconstituer le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Seulement 18 % de notre APD sont aujourd'hui tournés vers les services sociaux de base ; cet effort est appelé à être massivement amplifié. Le présent projet de budget affecte près de 1 milliard d'euros au Fonds vert pour le climat, afin de permettre à la France de tenir, à la dernière minute, la promesse formulée par Emmanuel Macron en 2019 au G7 de Biarritz d'abonder ce fonds de 1,5 milliard d'euros sur la période 2019-2023. C'est un pas en avant ; il faudra poursuivre sur cette lancée. COP après COP, les discussions achoppent sur la solidarité des pays industrialisés avec les pays en développement. Nous nous apprêtons enfin, en 2023, à tenir la promesse de 100 milliards par an faite à Copenhague en 2009.

et Proparco, afin d'éviter, comme nous avons failli le faire à Kahuzi-Biega en République démocratique du Congo (RDC), de nous rendre complices d'atrocités, et en continuant de plaider pour que notre aide publique prenne davantage la forme de dons, priorise les pays cibles, les services sociaux de base, la lutte contre le réchauffement climatique et respecte les populations locales, notamment les peuples autochtones. La

Vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur spécial, cette mission se compose de deux programmes : le programme 110, « Aide économique et financière au développement », porté par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et le programme 209, « Solidarité à l'égard des pays en développement », qui relève du Quai d'Orsay.

Avec ces moyens supplémentaires, le Quai d'Orsay va pouvoir poursuivre deux objectifs majeurs : la participation de la France à la gestion des enjeux globaux et sa contribution à la réduction des fractures qui déstabilisent le monde. concerne les enjeux globaux, la France entend continuer de contribuer activement à la définition et à la mise en oeuvre des réponses internationales à leur apporter. Évoquons d'abord le climat, défi absolu comme l'a montré la COP27 qui s'est achevée il y a quelques jours. La France devrait y consacrer 6 milliards d'euros par an sur la période 2021-2025, dont un tiers pour l'adaptation au changement climatique. Dans le cadre de cet effort, la France a augmenté massivement sa contribution au Fonds pour l'environnement mondial, passant de 217 millions à près de 300 millions d'euros par an sur le prochain cycle 2023-2026.

En outre, alors que se tiendra dans quelques jours la COP15 consacrée à la biodiversité à Montréal, la France souhaite renforcer sa mobilisation pour la protection de la nature. D'ici à 2030, 30 % de l'ensemble des financements bilatéraux français pour le climat auront aussi un impact bénéfique sur la biodiversité : le Président de la République s'y est engagé lors du de janvier 2021. Je signale, enfin, que la deuxième reconstitution du Fonds vert pour le climat interviendra en 2023. Une nouvelle hausse de notre contribution permettrait de préserver le rang de la France et de marquer la priorité donnée à l'action climatique. Des moyens ont d'ores et déjà été prévus sur le programme 110.

ou dans un cadre bilatéral, principalement en Afrique. Sur ce point, je signale que la nouvelle contribution française au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme s'élève pour 2023-2025 à 1,6 milliard soit une hausse de 23 % par rapport à 2019. Pour ce qui a trait à l'alimentation, le problème de la faim, qui touche 10 % de la population mondiale, est aggravé par l'invasion de l'Ukraine. En 2022, 205 millions de personnes seraient en situation de crise alimentaire dans quarante-cinq pays, en particulier en Afrique de l'Ouest. Afin de répondre la France compte mobiliser en 2023 des moyens supplémentaires, le canal de l'aide alimentaire programmée, laquelle passerait de 118 millions d'euros en 2022 à 160 millions d'euros en 2023. Nous souhaitons également renouveler notre contribution à l'initiative (Farm).

est aujourd'hui un enjeu majeur. Notre aide humanitaire pourrait atteindre 642 millions d'euros au travers de trois canaux principaux : outre l'enveloppe d'aide alimentaire programmée et le soutien

notre diplomatie aura les moyens de ses ambitions. Ce budget reflète les fortes attentes à l'égard de notre diplomatie, mais aussi la confiance que lui témoignent nos plus hautes autorités. C'est une confiance qui doit

notre politique de développement constitue une véritable priorité politique du Gouvernement. En cinq ans, nous avons doublé les crédits de la mission « Aide publique au développement ». Cela représente une hausse historique de 2,5 milliards d'euros. Surtout, nous allons tenir l'engagement pris par le Président de la République en 2018, en consacrant 0,55 % de notre revenu national à l'APD en 2022. Comme vous le voyez, nous investissons donc plus, mais surtout nous investissons mieux. Notre APD comprend désormais davantage d'aides bilatérales et de dons. Ces dons sont dirigés vers les pays les plus vulnérables- particulièrement les pays du continent africain -et ils sont concentrés sur les secteurs du développement humain, tels que l'éducation et la santé. Nous investissons aussi mieux. En renforçant l'expertise technique, nous renforçons en même temps les liens humains entre notre pays et les pays partenaires. En donnant plus de moyens à nos ambassades, nous leur permettons de promouvoir des projets concrets et visibles, au plus près des besoins des populations. Depuis cinq ans, nous ne faisons pas seulement plus et mieux, nous employons surtout une nouvelle méthode. Désormais, nous veillons à travailler avec les pays du Sud pour soutenir leurs initiatives et répondre à leurs besoins. Il s'agit pour nous d'accompagner ces pays pour relever ensemble les grands défis globaux qu'évoquait Mme la ministre Colonna. Je pense, par exemple, à ce que nous avons fait durant la pandémie pour la vaccination des pays du Sud. Nous avons su nous réunir, en Européens, pour appuyer le renforcement des capacités africaines de production de vaccins.

Nous demandons à chacun de nos opérateurs, notamment à l'Agence française de développement, de mettre en oeuvre cette approche. Pour chaque Français, cette politique de développement doit être une fierté. Elle fait rayonner nos idéaux de solidarité. au-delà de cette fierté, mesdames et messieurs les sénateurs, cette politique de développement nous permet directement de protéger les Français et leurs intérêts. Nous vivons dans un monde Lorsque nous renforçons les systèmes de santé des pays du Sud, c'est la santé de nos concitoyens que nous protégeons. Lorsque nous protégeons les forêts du bassin du Congo, c'est notre climat aussi que nous préservons. Investir dans le développement, trouver de nouveaux alliés est la meilleure manière de faire peser peser notre vision du monde : celle de la coopération, du multilatéralisme, du respect de la souveraineté de chacun. Cette vision, c'est celle de la France, c'est celle de l'Europe, mais c'est aussi la vision que le

Il nous paraît ainsi logique qu'une mission augmentant significativement ses moyens participe également à cette volonté de maîtrise de la dépense publique. C'est la raison pour laquelle la commission des finances vous propose un amendement visant à réduire de 200 millions d'euros les crédits dédiés à l'aide publique

cela passera par pertes et profits pour des problèmes internes à un parti politique

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

d'autant qu'ils sont les plus touchés par les chocs économiques, climatiques ou autres. Pour toutes ces raisons, nous proposons de doubler les crédits supplémentaires accordés au compte de bonification, ce qui permettrait de réduire le taux de bonification des DTS.

dotée de 130 millions d'euros en 2023. Cet amendement vise à augmenter le montant de l'encours de prêts à taux zéro accordés par la Banque de France, qui bénéficient de la garantie de l'État en vertu des dispositions de la loi de finances pour 2022. En premier lieu, le montant de l'encours des prêts concessionnels

aux pays les plus pauvres. Vous le savez, le Président de la République avait lancé cette idée en 2021, lors du sommet sur le financement des économies africaines (SFEA). Au-delà de l'objectif des 20 % fixé par le G20, la France s'est engagée à réallouer jusqu'à 30 % des DTS. Dans le cadre du budget 2022-2023, la France y contribue à hauteur de 5 milliards d'euros, ce qui correspond à notre engagement de 20 %, et nous sommes en discussion avec le FMI pour voir comment nous Les besoins de bonification qui accompagnent cette réallocation sont bien pris en compte dans les crédits du programme 110, avec 40 millions d'euros consacrés à la FRPC et au Fonds mondial pour la résilience. Ces montants sont jugés suffisants par le FMI. Enfin, une telle réduction des crédits du programme 209 serait en totale contradiction avec la priorité que nous souhaitons tous accorder à notre action sous forme de dons. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

vont prioritairement vers les pays les plus pauvres- ceux qui en ont le plus besoin -, profitant ainsi aux populations les plus vulnérables et aux secteurs sociaux qui constituent la base du développement. La France est l'un des pays qui orientent le moins leur aide vers les services sociaux de base.

Il est vrai qu'aucun indicateur ne permet actuellement de rendre compte de la part des prêts et des dons alloués aux 19 pays prioritaires pour notre aide tant bilatérale que multilatérale, de manière générale. Cela s'explique par des difficultés inhérentes à la mesure de l'APD.

vous voulez, madame la ministre, modifier la présidence de la commission indépendante chargée d'évaluer l'efficacité et la destination de l'aide publique française pour placer ladite commission sous la présidence du Premier président de la Cour des comptes. Vous invoquez la difficulté, au regard de la composition de cette commission, de choisir un président,

deux observations, l'une sur la forme et l'autre sur le fond. Sur la forme, d'abord : il est évident que la manière dont le Gouvernement a procédé, avec du reste beaucoup de gêne,

lors de mon intervention liminaire, mais, selon nous, la loi du 4 août 2021 aurait dû être l'occasion de placer l'objectif de l'enregistrement des naissances et de la mise en place d'états civils fiables au rang des priorités de la politique de développement de la France.

devrait être l'occasion pour le Gouvernement de rendre compte des actions de la France en faveur de la promotion de la constitution d'états civils fiables, ainsi que de l'enregistrement des naissances et de la délivrance d'actes de naissance.

accroître la mobilisation internationale en faveur de l'état civil ; renforcer cette prise en compte dans l'aide publique au développement ; obtenir une meilleure communication sur les enjeux en la matière. Ces trois indicateurs font l'objet d'un rapport tous les deux ans et le premier de ces rapports doit être publié d'ici au mois de juin 2023.